La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 20 juin 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. La parole est à M. Patrick Kanner, pour un rappel au règlement. Madame la présidente, monsieur le secrétaire après le mouvement qui touche le personnel urgentiste depuis de très nombreuses semaines dans nos hôpitaux, ce sont les sapeurs-pompiers qui se mobilisent aujourd'hui avec un préavis de grève s'étendant du 26 juin au 31 août, tout en maintenant bien sûr leurs prestations pour le grand public. représentant 85 % des personnels ont prévu de se mobiliser ces prochains mois pour alerter sur un service de secours qui est malade- permettez-moi ce raccourci. Ces personnels doivent répondre à une sursollicitation, malgré une baisse d'effectifs et de moyens, en assumant de plus en plus des missions qui ne relèvent pas de leurs compétences, chacun des élus locaux ici peut en témoigner. Ils subissent de plein fouet les manquements de l'État, mais aussi des difficultés au sein de chaque département. Monsieur le secrétaire d'État, alors que le Gouvernement s'enorgueillit de poser les bases d'un « nouveau contrat social »- je reprends l'expression -avec la fonction publique- et que nous contestons, vous l'avez compris -, cet épisode nous fait craindre que le compte n'y soit pas. Le préavis transmis au ministre de l'intérieur rappelle notamment les problématiques liées à la sécurité des sapeurs-pompiers, délaissée par le Gouvernement et dont le Sénat s'est saisi par le biais d'une mission d'information À cet égard, je salue mon collègue Loïc Hervé. collègue Loïc Hervé. Ces sapeurs-pompiers demandent le retrait de votre projet de loi de transformation de la fonction publique, débattu aujourd'hui dans cet hémicycle, car celui-ci fait porter, comme nous le pensons aussi, un risque majeur de fragilisation du service public au travers de la fonction publique. Nous ne doutons pas que vous ne donniez pas suite à cette demande, qui nous semblerait pourtant légitime. Ce rappel au règlement est l'occasion pour moi et pour le groupe socialiste et républicain de vous interpeller sur la nécessaire réponse qu'il faudrait apporter à cette profession qui souffre. Monsieur le secrétaire d'État, que comptez-vous faire ? Cela fait tant d'années que les pompiers expriment des doléances ! Ils sont les témoins privilégiés des fractures sociales de notre société, il est temps, plus que temps, de les écouter. Le Gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure de cette situation. Nous regrettons la crispation du dialogue social avec une profession

Mme Fabienne Keller a fait connaître à la présidence qu'elle se démettait de son mandat de sénateur du Bas-Rhin à compter du 23 juin 2019, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, elle est remplacée par Mme Esther Sittler, dont le mandat de sénatrice a commencé le 24 juin 2019, à zéro heure. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement 13 de la Constitution sont parvenues à l'adoption de textes communs. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, Didier Marie et moi-même avons rendu un rapport pour « donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », rapport qui a nécessité 8 mois de travaux, 2 déplacements et l'audition de 104 parties prenantes. Ce rapport a été adopté à l'unanimité par la commission des lois. Globalement, la situation s'améliore et nous pouvons nous en féliciter : le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est passé de 3,74 % en 2006 à 5,61 % aujourd'hui. Toutefois, nous avons constaté trois principales difficultés. Premièrement, seul le versant territorial respecte ses obligations. L'État est en retard avec 4,65 % d'agents handicapés- et seulement 3,38 % dans les services du Premier ministre. Deuxièmement, les actions menées reposent souvent sur l'engagement personnel de certains élus, managers ou agents. Elles sont mises à mal lorsque ces locomotives quittent leurs fonctions. enfin, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, connaît une situation financière très préoccupante, après avoir accumulé 230 millions d'euros de déficit entre 2015 et 2018. Il a dû baisser ses aides aux agents handicapés, ce qui n'est pas satisfaisant. Face à ces constats, le projet de loi initial restait en retrait. Il se limitait à confirmer des interprétations déjà en vigueur, comme l'a souligné le Conseil d'État. Un seul dispositif nous paraît novateur : la création d'un détachement pour favoriser la promotion des agents porteurs de handicap. notre initiative, la commission des lois a adopté six amendements pour mieux intégrer les personnes handicapées dans la fonction publique. Certains semblent recevoir l'approbation du Gouvernement, comme la généralisation des référents handicap, le droit à la portabilité des aménagements de poste ou la possibilité de titulariser, à titre expérimental, un apprenti handicapé à l'issue de son contrat d'apprentissage. Toutefois, monsieur le secrétaire d'État, le compte n'y est pas. Vous proposez plusieurs amendements de suppression, précisant que le Gouvernement a déjà porté le budget du FIPHFP à 130 millions d'euros après la loi Pénicaud de septembre 2018. Or cette somme, selon nous, permettrait uniquement de couvrir les interventions du fonds, non ses frais de gestion. Il lui faudrait au moins 20 millions de plus, comme nous l'avons démontré dans notre rapport. Devant la commission des lois, vous avez indiqué que vous souhaitiez une certaine harmonisation entre le secteur public et le secteur privé.

À rebours de votre position de principe, vous souhaitez d'ailleurs supprimer des dispositions de la commission qui respectent votre volonté d'harmoniser le secteur privé et le secteur public. Je pense, par exemple, à la règle de l'arrondi à l'unité supérieure, qui rapporterait 13 millions d'euros par an au FIPHFP, ou au meilleur encadrement des maintiens dans l'emploi.

Vous l'aurez compris, monsieur le secrétaire d'État, nous souhaitons des avancées réelles et concrètes pour l'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique. Au cours de ce débat, nous espérons vous convaincre

Depuis la loi du 11 février 2005, les employeurs ont consenti de nombreux efforts pour relever le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique, qui est passé de 3,74 % à 5,61 %. Il faut souligner que, chaque année, les administrations recrutent plus de 30 000 agents handicapés, soit deux fois plus qu'en 2019. Pour autant, les objectifs assignés en 2005 ne sont que partiellement atteints et le système de promotion du handicap dans la fonction publique est aujourd'hui à un tournant, voire à bout de souffle. le versant territorial respecte son obligation d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés, sachant que, dans la fonction publique territoriale, il existe bien évidemment des écarts d'une collectivité à l'autre et qu'il ne faudra pas relâcher les efforts. Pour ce qui concerne l'État, il est en retard, avec un taux d'emploi de 4,65 %. Certains ministères, voire certains services, notamment ceux du Premier ministre, cela a été souligné, sont particulièrement en retard nous souhaiterions que l'État montre la voie, qu'il soit l'éclaireur et qu'il puisse dans un délai extrêmement rapide- deux ans

les services de l'État manquaient de coordination. Se pose la question de la déconcentration des moyens dévolus au handicap dans la fonction publique d'État. Le second sujet fondamental, c'est effectivement celui du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Après avoir contribué à une élévation du nombre de travailleurs handicapés dans les trois fonctions publiques, a malheureusement été contraint de réduire drastiquement le montant de ses aides, qui ont baissé de 30 % entre 2014 et 2018, victime au final de son succès. Il faut conclure, mon cher collègue. Vous avez épuisé votre temps de parole. Nous vous demandons de regarder avec beaucoup d'attention- c'est l'objet du présent projet de loi -la mise en oeuvre d'une expérimentation de réforme globale du modèle de financement du FIPHFP. La parole est à M. Philippe Mouiller, d'essayer de respecter le temps qui lui est imparti.

c'est qu'un certain nombre des dispositions que vous avez adoptées, au-delà de leur intérêt propre, ne soient contradictoires avec cette volonté de faire converger les secteurs public et privé en matière de handicap.

permettra une montée en puissance de la contribution du ministère de l'éducation nationale et donc de garantir l'alimentation du FIPHFP, indépendamment des efforts faits en matière d'accueil des personnes en situation de handicap, à hauteur de 130 millions

des engagements et des efforts à fournir en matière d'accueil. Enfin, je termine sur ce que l'on pourrait qualifier de divergence, laquelle peut, à mon avis, être surmontée.

que nous considérons, à la commission des lois, que le compte n'y est paset que nous ne pouvons nous contenter de vous faire crédit de vos bonnes intentions. Vous connaissez les chiffres comme nous les connaissons. En 2014, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique avait un budget de 181 millions d'euros. Il est

qui avons créé ce fonds. Vous nous dites : « Il faut attendre. » Non, n'attendons surtout pas, ne ratons pas l'occasion du prochain budget de l'État pour amorcer un redressement Vous proposez 130 millions ; nous vous disons que 150 millions d'euros, c'est encore beaucoup moins qu'il y a cinq ans et c'est nécessaire. Cette évaluation n'est pas sortie de notre chapeau, elle résulte d'un travail pluraliste mené par M. Marie et Mme Di Folco, dont chacun, y compris vous-même, a salué le sérieux. a salué le sérieux. Pour assurer la pérennité des financements à un haut niveau, il est absolument indispensable de modifier le système de prélèvement. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce système de bonus-malus.

pour mettre en oeuvre un dispositif qui sera plus efficace pour les personnes handicapées ! C'est la raison pour laquelle, au moment d'aborder l'examen de ces amendements, je tiens à vous dire très solennellement

lequel vous voudriez rapprocher, sans les fusionner, le fonds pour le secteur privé et le fonds pour le secteur public ne nous paraît pas recevable, et ce pour une raison très simple : les modalités de recrutement, le déroulement des carrières et même les métiers sont différents entre le secteur privé et le secteur public.

jouerait en défaveur des financements spécifiques pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Cet argument ne saurait retarder ce travail devant nous permettre de franchir un palier dans l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. C'est ce que le Sénat vous demande. Vous dites que nous sommes d'accord sur les objectifs ; eh bien, je souhaite maintenant que nous soyons aussi d'accord sur les moyens

qui n'est pas acceptable, même si l'on annonce une nouvelle fois un code de la fonction publique ; la limitation à cinq ans de la prise en compte des maintiens dans l'emploi dans le calcul du taux d'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ne pas avantager les employeurs qui « fabriquent » du handicap ; la règle de l'arrondi à l'inférieur, qui permettrait d'augmenter les contributions au FIPHFP de 13 millions d'euros ; la modernisation du conventionnement entre le FIPHFP et les employeurs publics, ayant notamment permis la publication des objectifs retenus et des résultats obtenus. Le Gouvernement accepte simplement de revoir la « tripartition » du FIPHFP entre les trois versants de la fonction publique, ce qui n'a jamais été appliqué. L'ambition du Gouvernement, au travers de cet amendement, est donc bien plus limitée que le rapport du Sénat, alors qu'il y a urgence à donner un nouveau souffle

de la commission ? Avec cet amendement, le Gouvernement souhaite supprimer une proposition du Sénat relative au handicap dans la fonction publique. Le système actuel du financement du FIPHFP connaît deux difficultés principales. Premièrement, ce fonds subit un effet de ciseaux : avec la progression du nombre d'agents handicapés, les ressources du fonds s'amenuisent alors que les besoins de financement augmentent. Ces dernières années, le fonds a réduit de 40 % le montant de ses conventions avec les employeurs publics, au détriment des agents en situation de handicap. Deuxièmement, le système actuel favorise les employeurs publics qui « créent » du handicap. Plus les agents sont exposés à des risques professionnels, plus ils sont reclassés, ce qui permet de réduire d'autant les contributions de leur employeur. un véritable effet pervers. Face à ces difficultés structurelles, le Gouvernement a prévu un « sparadrap », c'est-à-dire des mesures ponctuelles pour stabiliser les ressources du fonds à 130 millions d'euros. Certaines mesures sont courageuses, comme la réduction des dérogations accordées par l'Assemblée nationale. ces dispositions sont insuffisantes pour régler l'effet de ciseaux constaté. Pis, elles ne répondent pas aux besoins du FIPHFP, que le Sénat a estimés à 150 millions d'euros. Dès lors, il est important de lancer une expérimentation pour refonder le modèle

pour valoriser les employeurs vertueux. Ce bonus-malus est également la seule manière de pénaliser les employeurs qui multiplient les retraites ou les licenciements pour inaptitude. Comment être contre cette solution de bon sens ?

réduction de 40 % du montant des conventions employeurs- ce sont les conventions que le fonds passe avec des employeurs publics pour obtenir de ceux-ci l'engagement de recruter des personnes handicapées et de les accompagner dans leur travail ; plafonnement des aides ponctuelles à 100 000 euros sur trois ans ; instauration d'un plancher de prise en charge, les dépenses de moins de 200 euros n'étant plus remboursées par le fonds

suppression des aides accordées pour assurer l'accessibilité des bâtiments. Il faut donner un coup d'arrêt à ce rétrécissement de la capacité d'action

le papa d'un jeune handicapé que je suis apprécie assez modérément l'instrumentalisation que certains échanges pourraient donner l'impression de développer. Ces sujets concernent un certain

par ce biais, d'aucune visibilité. En outre, le recours à la loi est nécessaire pour prévoir les conditions dans lesquelles des personnes handicapées pourraient déposer leur curriculum vitae

pas l'auteur : le rapport de Catherine Di Folco et Didier Marie, c'est 8 mois de travail, c'est 104 auditions, c'est une adoption à l'unanimité par la commission des lois du Sénat. C'est donc un travail sérieux, et c'est une approche du handicap dans la fonction publique qui se veut la plus universelle et la plus bienveillante possible.

à cette partie du texte

Comment expliquer que des agents publics répondant à un besoin permanent, indispensables au bon fonctionnement de l'éducation nationale, soient laissés dans une précarité absolue ? C'est bien le premier enjeu d'un statut de fonctionnaires pour les AESH : la sortie de la

les établissements sont recruteurs, ou encore en fonction des académies et des directions desdits établissements. Le recrutement se fait, en dépit du bon sens, à temps partiel et à durée déterminée, ce qui entraîne des rémunérations particulièrement faibles et une imprévisibilité

Fonctionnariser les AESH constituerait une solution juste socialement pour ces derniers et une garantie pour qu'ils soient affectés en amont de la rentrée scolaire. Par ailleurs, il faut relever que, en l'absence de cadre, les AESH ont bien du mal

du service public d'éducation. Le ministre de l'éducation nationale a pointé, à juste titre, les difficultés qu'il avait à recruter des AESH. Au vu du tableau que je viens de dépeindre, cela n'est guère étonnant ; et ce n'est pas en assouplissant les conditions de recrutement,

d'évoquer un sujet important, et elles nous permettront d'entendre le Gouvernement sur ce point. Aujourd'hui, les AESH gagnent en moyenne 700 euros par mois, sur la base de contrats précaires seuls 2 % d'entre eux travaillent à temps plein. Le Gouvernement a pris plusieurs engagements, notamment de porter à 30 % la proportion d'AESH à temps plein d'ici à la rentrée prochaine, ou encore de permettre l'octroi d'un CDI lorsqu'un AESH a obtenu deux CDD de trois ans. Nous attendons que le Gouvernement nous détaille ses engagements et, surtout, qu'il les tienne !

particulièrement, les questions que vous évoquez, à l'issue d'une large concertation avec les partenaires sociaux, le ministère a adopté un nouveau cadre de gestion de ses agents. Il s'agit d'un des leviers essentiels du saut qualitatif annoncé, lequel est nécessaire pour construire une école inclusive et transformer durablement le dispositif d'accompagnement. le dispositif d'accompagnement. Ce nouveau cadre pose les fondements d'une gestion pérenne et valorisante des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Il définit des mesures de nature à consolider leur place dans la communauté éducative, en améliorant à la fois leur gestion administrative et leurs conditions d'exercice, avec l'allongement de la durée des contrats, l'accroissement de la quotité travaillée et la meilleure prise en compte, en rémunération, des activités connexes à l'accompagnement des élèves. Les travaux dont il s'agit ont vocation à se poursuivre pour renforcer ces acquis fondamentaux. Ils s'appuient sur une réflexion aboutie.

conduirait,, à appliquer aux mêmes AESH des règles de gestion potentiellement moins favorables que les dispositions définies dans le nouveau cadre de gestion que le ministre de l'éducation nationale met en place. En particulier, la gestion d'un corps impliquant d'éventuelles mobilités à l'échelle académique ou départementale,

tous les nouveaux AESH seront recrutés au 20 août prochain. Entre cette date et celle de la rentrée scolaire, ils bénéficieront

lors de leur recrutement. Des efforts doivent être réalisés pour l'adaptation des épreuves des concours et des examens de la fonction publique, comme pour la sensibilisation des personnels chargés des ressources humaines. Surtout, le nombre de postes ouverts aux handicapés doit La mission d'information sur la politique de l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, menée par Catherine Di Folco et Didier Marie, à laquelle notre rapporteur, Loïc Hervé, a d'ailleurs fait référence, a permis de chiffrer à 280 760 le nombre de travailleuses et de travailleurs handicapés

dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Je signale que cet effort, quoique insuffisant, est plus important dans les collectivités territoriales, puisque le taux de fonctionnaires handicapés

des agents qui y concourent, au profit d'une contractualisation à outrance. Nous continuons de nous y opposer et de défendre l'ensemble des fonctionnaires, y compris, bien entendu, les fonctionnaires handicapés.

professionnel des personnes en situation de handicap engagées dans la fonction publique. Il entend, de plus, faciliter la mise en oeuvre d'aménagements en leur faveur lors du déroulement des épreuves des concours et examens. Si les intentions sont louables, le système d'aide aux travailleurs handicapés est à bout de souffle, comme le dénonce d'ailleurs un récent rapport de la commission des lois du Sénat. Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, destiné à financer des actions pour favoriser l'emploi de ces personnes et leur insertion professionnelle, est en grande difficulté financière ses aides ont ainsi baissé de 30 % entre 2014 et 2018. Les personnes handicapées, souffrant déjà d'invisibilisation et de stigmatisation en France, sont pourtant des acteurs indispensables pour notre administration, qui doit refléter notre société dans toute sa diversité. Aussi, nous aurions souhaité que le recrutement par voie contractuelle soit assoupli, afin de multiplier les titularisations de ces agents. Il n'en est rien dans ce projet de loi.

En 2019, nous sommes malheureusement toujours en deçà de cette obligation légale, notamment dans la fonction publique d'État, dans laquelle les personnes handicapées représentent seulement 4,65 % des effectifs. Le Gouvernement n'a manifestement pas pris en compte ces appels à l'aide et a manqué, une fois de plus, de la volonté de mieux faire, prouvant ainsi que la protection des plus vulnérables n'était pas sa priorité. L'amendement

Cartron. Cet amendement vise à suggérer une nouvelle rédaction de la disposition permettant à tout agent public de consulter un référent handicap,

actuellement rédigé, l'alinéa 6 se borne en effet à évoquer les seules conditions d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Or je persiste à croire que cette sobriété légistique n'est pas si raisonnable qu'il y paraît. Mes chers collègues, décrire un handicap, c'est définir les moyens de l'appréhender et, par là même, organiser les conditions de son acceptabilité sociale. Parler de « maintien » et d'« insertion », c'est déjà imprimer dans la loi un présupposé inégalitaire. Être traité en handicapé, voilà bien le premier des handicaps ! Nos textes de loi doivent être soucieux de ces formules de langage : en aucune façon, le « maintien » dans un emploi ne saurait être vécu comme une forme d'accomplissement professionnel. Nous préférons, en ce sens, voir reconnaître au référent un rôle plus dynamique et plus positif, corrélé, par nature, à la possibilité pour l'agent en situation de handicap d'accéder à des fonctions de niveau supérieur. Par ailleurs, il nous semblait opportun de préciser que le référent handicap devait oeuvrer concomitamment à la sensibilisation de l'ensemble des agents

Longeot. Beaucoup reste à faire pour que les personnes handicapées puissent s'intégrer convenablement et durablement au sein du marché du travail. J'en veux pour preuve que leur taux de chômage reste deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Au sein de la fonction publique, de réels progrès ont été constatés ces dernières années, notamment à la suite de l'introduction de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés : entre 2006 et 2018, le taux d'emploi légal des personnes handicapées est passé de 3,74 % à 5,61 %. Chaque année, ce sont ainsi plus de 30 000 travailleurs handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique, soit deux fois plus qu'en 2009. Ces derniers rencontrent toutefois de véritables obstacles, identifiés dans l'excellent rapport de nos collègues Catherine Di Folco et Didier Marie relatif au handicap dans la fonction publique.

ne bénéficient aujourd'hui d'aucune garantie statutaire, ce qui peut parfois freiner l'accompagnement des agents handicapés et empêcher certains d'entre eux de trouver un emploi pérenne au sein de la fonction publique.

Le tuteur complétera utilement le rôle du référent déontologue chargé d'impulser la politique du handicap dans chaque administration. La commission y est favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

de la commission ? Notre définition du droit à la portabilité nous paraît plus concrète et plus opérationnelle. Nous notons toutefois que le Gouvernement accepte de reconnaître ce droit, ce qui constitue une avancée et met fin à des situations illogiques. L'agent conservera désormais ses aménagements de poste, adaptés à son handicap, lorsqu'il changera d'employeur. Le Gouvernement souhaite supprimer la consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs au handicap dans la fonction publique, quand les représentants des personnes en situation de handicap ont pourtant besoin d'être

le nombre de personnalités qualifiées nommées respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement s'est opposé à ce rééquilibrage au profit du Parlement, arguant de la nécessité de maintenir un équilibre entre les nominations relevant du Parlement et celles qui reviennent au Gouvernement. Pourtant, même dans cette configuration, les personnalités qualifiées nommées par les présidents des deux assemblées étaient minoritaires, au nombre de six dans un collège comptant treize membres. Nous proposons, par cet amendement, de rétablir cette composition, cohérente avec notre volonté de rehausser les droits du Parlement.

pour renforcer les contrôles déontologiques, tout en rappelant le droit, pour les fonctionnaires, d'avoir des expériences dans le privé. Nous avons notamment amélioré le suivi des réserves de la HATVP et renforcé le contrôle du rétropantouflage. Sur l'initiative du groupe socialiste et républicain, nous avons également généralisé les contrôles sur les collaborateurs du Président de la République et des cabinets ministériels. L'article 16, que nous abordons à présent, concerne l'organisation même de la Haute Autorité. Il est question non plus uniquement du contrôle du pantouflage des agents publics, mais, plus largement, du contrôle de la déontologie dans la sphère publique, incluant les membres du Gouvernement, les élus et les membres des autorités administratives indépendantes. Sur le fond, je vous propose d'en rester au texte de la commission et de refuser que le Gouvernement désigne deux membres supplémentaires au sein de la HATVP. De même, je ne suis pas favorable à la création d'une formation restreinte ou à la possibilité, pour le supérieur hiérarchique, de siéger au sein de la Haute Autorité, même avec une voix consultative. À la différence de la commission de déontologie, la Haute Autorité est une autorité administrative indépendante et rien ne doit laisser croire que le Gouvernement

La position de la commission me semble plus équilibrée : la HATVP comporterait onze membres, dont six magistrats, quatre membres désignés par le Parlement conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution et un président désigné par le Président de la République.

HATVP comptera donc onze membres, dont quatre nommés par le Parlement et un seul- le président -nommé par l'exécutif. En outre, l'adoption de l'amendement n° 144 rectifié rendrait plus difficile l'application du principe de la parité à la HATVP, qui sera

Le Gouvernement souhaite désigner deux représentants au sein du collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce que la commission a refusé à l'unanimité. En effet, le Gouvernement nomme déjà le président de la HATVP, qui dispose de larges pouvoirs, notamment en matière d'autosaisine.

Je préfère les nominations décidées par le Parlement, après audition publique des intéressés. En outre, l'Agence française anticorruption est un service rattaché au ministère de la justice ; sa présence pourrait donc renforcer l'exécutif, ce que la commission ne souhaite pas. Avis défavorable.

La HATVP pourra gérer l'afflux de dossiers en jouant sur l'organisation de ses réunions. La CNIL, par exemple, que j'évoquais à demi-mot, fonctionne avec une partie A donnant lieu à délibérations et une partie B donnant lieu à un vote plus global et à délibérations uniquement à la demande de l'un des commissaires.

aux réunions de la Haute Autorité. Notre avis est défavorable, car cela remettrait en cause, au moins dans les apparences, l'impartialité de la Haute Autorité, qui reste une autorité administrative indépendante. En outre, le VIII de l'article 25 de la loi Le Pors de 1983 permet déjà à la HATVP d'obtenir des informations en amont de ses réunions auprès de l'autorité hiérarchique ou de l'autorité de nomination. que les rapporteurs de la HATVP sont, en l'état du droit, des magistrats administratifs, financiers ou judiciaires. Ils préparent les dossiers les plus importants avant que ceux-ci ne soient soumis aux membres du collège.

mes auditions ; mais le président de la HATVP m'a convaincu qu'il était préférable d'en rester au droit en vigueur, car il pense pouvoir gérer le volume des affaires avec le vivier actuel de rapporteurs. Il nous semble difficile pour un fonctionnaire de l'État d'instruire le dossier d'un de ses collègues.

de Belenet propose que l'autorité hiérarchique ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que le référent déontologue dont relève l'intéressé, puissent, sans voix délibérative,

la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna -les dispositions prévues à l'article 16 en matière de transparence de la vie politique. En effet, l'organisation propre des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est fixée exclusivement par les lois organiques statutaires, y compris dans ce domaine, contrairement aux règles en vigueur à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, territoires régis par le principe de l'identité législative. Comme l'a déterminé le Conseil d'État dans sa décision d'assemblée du 9 février 1990 portant sur les élections municipales à Lifou, il ne suffit pas qu'un nouveau texte modifie un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable. En conséquence, dès lors que le projet de loi modifie la composition

Mes chers collègues, je suis particulièrement heureuse de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de parlementaires irlandais, conduite par M. Neale Richmond, sénateur et président du groupe interparlementaire d'amitié Irlande-France. La délégation est accompagnée par Mme Françoise Laborde, présidente du groupe d'amitié France-Irlande. La relation ancienne d'amitié qu'entretiennent l'Irlande et la France est plus que jamais nécessaire aujourd'hui, alors que le Royaume-Uni, partenaire économique majeur de nos deux pays, a décidé de quitter l'Union européenne. Après avoir échangé avec les membres du groupe d'amitié France-Irlande du Sénat et s'être entretenue avec des membres de la commission des affaires économiques pour évoquer les nombreux sujets sur lesquels nos pays ont un intérêt partagé, la délégation sera reçue demain à l'Assemblée nationale. Nous espérons que ce séjour à Paris sera fructueux et souhaitons à nos amis irlandais la bienvenue au Sénat français. ! Nous

Nous proposons de renforcer la diffusion de la culture déontologique en demandant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de publier annuellement une synthèse de ses avis et conseils en matière de déontologie.

d'un amendement de clarification, puisque les receveurs publics sont des agents de l'État, payés par l'État. La possibilité de leur verser une indemnité de conseil suscite chaque année des discussions au sein d'un assez grand nombre de collectivités

L'amendement présenté par M. Delahaye vise à supprimer l'indemnité de conseil que peuvent percevoir les agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État au titre

en proposant que le non-respect de l'engagement à servir l'État pour une durée minimale de dix ans soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire. Les élèves fonctionnaires sont rémunérés par l'État dès leur admission, en contrepartie de quoi ils s'engagent à servir l'État pendant dix années. Si la règle des dix ans n'est pas respectée, les élèves sont censés rembourser une partie des traitements perçus pendant leur formation. Toutefois, cette règle n'est pas suffisamment dissuasive.

L'encadrement, voire l'interdiction du pantouflage est ancienne, puisqu'elle fut introduite dès 1919, voilà donc un siècle ; elle a été constamment réaffirmée depuis lors. Pourtant, cette interdiction n'est absolument pas suivie d'effets. Il se dit dans certains milieux que le plus gros employeur d'inspecteurs généraux des finances publiques est non pas Bercy, mais BNP Paribas ... La violation de cet interdit légal, mais aussi éthique, est monnaie courante, accentuée par la quasi-certitude d'une totale impunité. Il s'agit désormais du déroulement normal de carrière, au point qu'il est naturel de voir figurer dans un curriculum vitae le passage dans un ministère, puis dans une entreprise- non sans lien avec ledit ministère

C'est pourquoi, reprenant une des préconisations du rapport de notre excellent collègue Pierre-Yves Collombat, nous proposons une mesure simple et radicale pour enrayer ce phénomène : interdire toute forme de pantouflage, sauf à être radié de la fonction publique en devant rembourser l'ensemble des frais engendrés par la formation.

en droit d'attendre des réponses du Gouvernement. Le principe est déjà clairement posé : les fonctionnaires qui partent avant d'avoir accompli leur obligation de servir doivent rembourser leurs frais de scolarité. La durée de l'obligation de servir varie toutefois d'un corps à l'autre : elle est de dix ans pour l'École nationale d'administration, de huit pour l'École des mines, Le pouvoir réglementaire a apporté de premières réponses en 2017, puis 2019, notamment en empêchant les départs pendant les quatre premières années de service. Un manque de transparence persiste toutefois. Il existe peu d'informations sur le sujet, et les dispositifs ne sont pas clairement coordonnés : le recouvrement de la pantoufle échoit, selon le cas, au ministère ou à l'école. Ainsi, les deux commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la haute fonction publique ont eu de nombreuses difficultés pour investiguer sur ce point. Je souhaite avancer sur ces sujets, mais cet amendement me pose problème. Il vise à systématiser le licenciement des fonctionnaires n'ayant pas remboursé la pantoufle, alors qu'il faudrait sans doute prendre en compte des cas spécifiques ; je pense en particulier à des problèmes de santé.

on est pendant quelques années à BNP Paribas ou à la Société générale, ensuite à la tête de la Banque de France, puis on repart. repart. À cha peu, comme disait ma grand-mère, on finira bien par faire les dix ans ... Et puis, quand on sera installé dans une banque à un bon niveau, ma foi, on pourra rembourser une partie de la pantoufle.

des allers-retours des gens qui ont des postes de responsabilité- les autres, ce n'est pas important. C'est cela qui pose problème pour notre démocratie ! Or, en la matière, je ne sens pas un enthousiasme considérable de la part du Gouvernement

La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

La République En Marche. Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Cette semaine, un épisode caniculaire intense et précoce s'abat sur l'Hexagone, avec des températures supérieures à quarante degrés et des ressentis encore plus élevés. Certes, des leçons ont été tirées du tragique été 2003. Aujourd'hui, l'ensemble des ministères et des administrations se sentent concernés et ont déjà pris des mesures de prévention, qu'il s'agisse du report des épreuves du brevet, des préconisations aux entreprises, notamment dans le BTP, ou encore du recours facilité à la circulation différenciée en cas de pollution. Pour autant, madame la ministre, à l'échelle de toute une population, les réflexes individuels et collectifs en matière de prévention ne sont pas encore automatisés, même dans l'hémicycle, où la cravate reste de mise pour mes collègues masculins ... Aussi, pourriez-vous nous détailler les principaux éléments du plan Canicule déclenché cette semaine qui concerne la prévention, notamment les publics spécifiquement ciblés par les messages de prévention, ainsi que les mesures de mobilisation prévues pour les services de santé en cas d'afflux dans les hôpitaux et dans le secteur des services à la personne ? Comment la cellule de veille est-elle déclinée ?

les associations sportives. Nous travaillons également avec toutes les associations de lutte contre la précarité pour augmenter le nombre de maraudes et élargir les plages d'ouverture des centres d'hébergement de jour.

bleus dans les Ehpad existent depuis 2003. Toutes les consignes sont très bien connues des personnels, et nous suivons chaque jour, les agences régionales de santé, les hôpitaux qui seraient en tension, de façon à pouvoir les accompagner. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de signal d'alerte des établissements de santé. La parole

en septembre dernier, célébrait ses quarante ans de programmation. Depuis 1978, cette édition a réussi à s'imposer comme l'un des journaux télévisés préférés des Français, attirant près de 600 000 spectateurs en moyenne tous les soirs, avec, régulièrement, des pics de 1,5 million de téléspectateurs, pour suivre l'actualité, principalement locale. Cette situation aurait pu durer, mais c'était sans compter sur l'annonce des nouvelles orientations stratégiques de France Télévisions. Officiellement, on parle non pas de suppression de programme, mais de transfert sur Franceinfo. Pourtant, la disparition de l'émission, telle que nous la connaissons tous, semble inévitable, monsieur le ministre. Rebaptisé, remodelé et repensé, le futur n'a, à ce jour, même pas l'assurance que l'ensemble des moyens alloués au soient redéployés. Et pour cause, si la nouvelle édition est toujours consacrée à « l'international, l'Europe, la politique nationale, l'économie, et l'environnement », le coup de projecteur quotidien qui était mis sur nos régions et nos territoires va s'éteindre et, avec lui, une certaine idée du service public. Dans le contexte de l'examen prochain du projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel, quel modèle souhaitez-vous défendre, monsieur le ministre ? Celui de la numérisation à tout prix et de la généralisation des chaînes d'infos à toute vitesse ? Ou serez-vous- vous connaissant, je n'en doute pas ! -à l'écoute des maires ruraux, qui ont lancé une pétition pour s'opposer à ce transfert, afin de maintenir une édition locale, proche de leur collectivité ? Écouterez-vous le CSE, le comité social et économique, de l'établissement, qui s'est opposé hier à l'unanimité à la décision de la direction de France Télévisions, pour défendre un programme audiovisuel regardé par des téléspectateurs, notamment des seniors, qui ne se servent pas des nouvelles sources d'information écouterez-vous les usagers-citoyens qui plébiscitent leurs programmes et qui, pour beaucoup d'entre eux, vous regardent aujourd'hui ? Monsieur le ministre, vous êtes le dernier recours, et nous sommes très nombreux à compter sur vous ! La parole

En ce qui concerne l'information et la proximité, il est nécessaire d'adapter les programmes à l'évolution des usages de nos compatriotes, notamment à l'utilisation du numérique, mais pas seulement.

La direction a souhaité aller plus loin dans la réorganisation des programmes en matière d'information, en sanctuarisant les deux rendez-vous sur France 3 et sur France 2 de milieu de journée et de fin d'après-midi,

pouvoir accompagner la direction de la chaîne dans la transformation de ses programmes au service d'une meilleure satisfaction des missions de service public, ... Il faut conclure ! ... notamment en matière d'information

la mobilisation qui a eu lieu ce week-end à Belfort montre à quel point un énième renoncement en matière industrielle est devenu inacceptable pour une très grande diversité de nos concitoyens, les syndicats des salariés, les organisations d'employeurs, ainsi que les élus de tous bords Le Gouvernement répète souhaiter diminuer le nombre de salariés concernés par le plan social. Mais ce qu'il faut, c'est que la puissance publique se redonne des leviers en matière industrielle pour construire une véritable transition énergétique. Or nous nous sommes dépossédés, un à un, de tous nos fleurons, au point que nos emplois, nos savoir-faire, notre souveraineté économique et énergétique sont aujourd'hui à la merci de dirigeants sans scrupules, pour lesquels l'accroissement des profits est la principale, pour ne pas dire l'unique boussole. General Electric s'est engagé à créer 1 000 emplois ; vous devez lui faire respecter ses engagements, monsieur le secrétaire d'État ! Au-delà, comptez-vous obtenir un moratoire sur les suppressions d'emplois industriels, notamment dans la filière de l'énergie, qui doit être accompagné d'un plan de développement, indispensable pour assurer une véritable transition énergétique ?

sur celle de l'industrie et des emplois industriels. Nous vivons, il est vrai, une période assez paradoxale. La France crée de l'emploi industriel, des usines sont ouvertes, des entreprises investissent, et c'est heureux pour l'ensemble de nos concitoyens. Malgré l'amélioration de la situation industrielle et de la compétitivité de notre pays, qui tient aussi évidemment à l'ensemble des mesures mises en oeuvre par le Gouvernement pour accompagner cette compétitivité, nous rencontrons des difficultés sur un certain nombre de sites.

aux représentants des organisations syndicales que l'ensemble de ses services et lui-même se tenaient à leur disposition pour les accompagner dans un dialogue qui soit le plus constructif possible. Il est évidemment temps

que le plan présenté par General Electric soit le prélude à une fermeture du site de Belfort. Il faut réagir alors ! Au contraire, nous voulons que les investissements sur le site lui permettent de bénéficier de la reprise du marché des turbines lorsque celle-ci adviendra.

Il y a encore beaucoup à faire, mais cela passera par un dialogue aussi constructif que possible entre les organisations syndicales, General Electric et le ministère de l'économie et des finances.

travers le pays, dans beaucoup de tribunaux, les greffières et les greffiers, chevilles ouvrières du système judiciaire français, sont en sous-effectif. Les exemples sont nombreux : au tribunal de grande instance de Valence, mais aussi dans bien d'autres endroits, leur trop petit nombre ne leur permet pas d'absorber la charge de travail qui leur incombe. Cette situation entraîne l'allongement considérable du délai de traitement des dossiers. En effet, lorsqu'une décision de justice est prise par un magistrat, elle nécessite la rédaction par un greffier ou une greffière d'une notification, qui la rend valable aux yeux de la loi. Aucun dossier ne peut avancer sans cela, et ce sont les plus fragiles qui en souffrent en premier lieu, notamment les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ainsi que les enfants. Plusieurs centaines de dossiers traités par le tribunal pour enfants de Valence sont en attente depuis des mois et s'accumulent. Or, pour intervenir auprès des familles et mettre en oeuvre les décisions de justice prises en faveur de la protection de l'enfant, et de la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ont besoin de ces notifications rédigées par les greffiers, sans quoi ils n'ont aucun mandat pour agir. À cause du manque de personnel dans le service public de la justice, ils sont dans l'incapacité d'oeuvrer

elle a un rapport avec l'enfance en danger, et nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état. Vous m'alertez sur les difficultés du tribunal pour enfants de Valence qui se sont fait jour vers le mois de janvier dernier, notamment en raison de l'augmentation considérable du nombre de mesures d'assistance éducative.

Au tribunal pour enfants de Valence, les mesures d'assistance éducative ont augmenté de 60 % en quatre ans. Pour faire face à cette situation, nous avons affecté un magistrat supplémentaire l'année dernière. Nous avons ainsi pris en compte les difficultés existantes. Toutefois, l'organisation du greffe n'a pas suivi. suivi. C'est la raison pour laquelle il a fallu travailler localement : la présidente du tribunal de grande instance a organisé des réunions au mois de mai dernier, et la notification des décisions par les greffiers a depuis lors repris. Cependant,

un emploi supplémentaire dans ce cadre-là. Enfin, deux greffiers supplémentaires arriveront au mois de septembre prochain. Nous espérons ainsi pouvoir assurer au tribunal pour enfants de Valence les conditions nécessaires à son fonctionnement. Plus généralement, pour ce qui concerne l'exécution des décisions

Depuis la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, l'État facture le coût d'intervention des forces de l'ordre sur les manifestations sportives, récréatives ou culturelles organisées par les associatifs, mais aussi par les collectivités. À la suite des attentats de 2015, les mesures de sûreté ont été renforcées et le montant des frais de sécurité a explosé. La circulaire Collomb du 15 mai 2018 a entériné cette hausse et mis en péril de nombreuses associations et manifestations. À titre d'exemple, le montant facturé aux Eurockéennes est passé de 30 000 euros en 2017 à 250 000 euros en 2018. Dans mon département, la Vienne, il est demandé à l'association Au Fil du Son, gérée par 100 bénévoles, entre 15 000 et 30 000 euros pour trois jours de festival, sachant que cette association n'est pas encore informée du montant Dans les faits, l'application de cette circulaire est aléatoire ; certains critères sont sujets à interprétation par les préfets. Les factures diffèrent selon les départements pour des manifestations identiques. Un rapport a souligné la nécessité de clarifier la loi et d'harmoniser les pratiques. Un nouveau fonds d'intervention a heureusement pris le relais du fonds d'urgence, mais sa dotation est modeste et son périmètre restreint. Il ne contribuera pas au remboursement des frais de sécurité. Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre, pour assurer la pérennité de ces manifestations, qui sont les forces vives de nos territoires ?

des manifestations diverses et variées, les manifestations sportives et culturelles, qui peuvent mailler notre territoire et dont chacun ici connaît l'importance. Le premier sujet, le renforcement des conditions de sécurité

Le second sujet est celui de la facturation par l'État du coût de l'intervention des forces de sécurité intérieure, dans le cadre d'échanges avec les préfets et les associations ou les organisateurs de ces manifestations,

Monsieur le ministre, merci de votre réponse, mais ce n'est pas aux associations de financer une mission régalienne, celle d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a un risque de voir disparaître de nombreuses associations et de nombreux spectacles sur nos territoires.

ministre de l'intérieur, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, la délinquance explose à Paris. Les chiffres sont catastrophiques : hausse de 8 % des vols avec violence, progression de 34 % des vols à la tire, 10 % des cambriolages, sans parler de la multiplication des rixes entre bandes rivales, souvent composées de mineurs, n'est-ce pas, madame Belloubet ? ... La mairie de Paris réclame plus d'effectifs, mais cela ne résout pas les difficultés. Il faut nommer les vrais problèmes pour trouver les vraies solutions. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de faire baisser les chiffres de la délinquance, alors qu'il n'y a plus de policiers pour se porter candidat à l'investigation ? C'est pourtant la seule solution de nature à boucler des enquêtes et à faire diminuer de façon spectaculaire ces chiffres. Ensuite, il faut souligner la responsabilité de Mme la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui, avant de se convertir aux vertus de la police municipale pour des raisons ridiculement électorales, a joué au pompier pyromane par son appel de bienvenue à Paris lancé aux migrants en 2015. Résultat : les chiffres de la préfecture de police nous le rappellent, plus de 45 % des personnes mises en cause dans ces nouvelles délinquances sont des migrants. La préfecture de police, dont je salue l'efficacité dans la nouvelle gestion de l'ordre public face à la crise des gilets jaunes, parle de « l'effet important des vagues migratoires » : c'est écrit dans le journal du 21 juin dernier. Monsieur le ministre, l'insécurité devient la préoccupation quotidienne des Parisiens. Des quartiers entiers sont désormais des zones de non-droit. Que comptez-vous faire contre cette déflagration de la délinquance ?

augmenté son taux d'élucidation, c'est-à-dire son activité. Il convient donc de saluer le courage et la détermination de nos policiers et de la préfecture de police de Paris. Tout à fait ! Pour répondre au phénomène que vous avez dénoncé, monsieur le sénateur, sachez que,

contre la délinquance. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que la lutte contre la délinquance à Paris restera notre priorité. Le préfet de police, Christophe Castaner et moi-même mettons tout en oeuvre pour que ce soit le cas.

en ligne une vidéo qui dénonce les conditions de vie des bêtes dans la ferme expérimentale de Sourches. Ce centre privé européen de recherches en nutrition animale et conduite d'élevage y mène des expérimentations, afin d'élaborer de tester les aliments pour animaux de la marque Sanders, leader français en nutrition animale et filiale du groupe Avril. L'association pointe du doigt l'utilisation de hublots implantés dans le ventre des vaches, afin de permettre un accès direct à leur estomac

que cette pratique était choquante, mais restait scientifiquement utile et ne faisait en rien souffrir les animaux, eu égard à l'absence de stress, même s'il faudrait mieux l'encadrer à l'avenir. l'INRA, saisie de cette affaire, rendra ses conclusions d'ici à 2025. Ce reportage sur la condition animale et la manière dont on traite les bêtes au nom du sacro-saint rendement est, hélas, loin d'être le premier. J'espère que la pétition que j'ai personnellement signée aura une incidence sur le devenir de ce centre de recherches, dont la cruauté dépasse l'entendement. Le législateur doit faire entendre sa voix pour que l'animal ne soit pas qu'un maillon commercial. Madame la secrétaire d'État, que pouvez-vous répondre aux Français choqués par cette nouvelle affaire d'animaux bafoués, ainsi qu'aux éleveurs qui sont l'élément clé de cette filière et qui découvrent, comme moi, cette pratique ?

d'une pratique de recherche sur les ruminants qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, avec comme objectif la réduction des antibiotiques et des émissions de nitrate et de méthane. Je ne crois pas Je ne crois pas que l'on puisse se satisfaire de cette pratique, même si elle est ancienne et menée à des fins scientifiques. La communauté scientifique a le devoir de recourir à des méthodes alternatives, telles que le rumen artificiel ou la modélisation des processus digestifs, avec pour objectif de ne plus opérer de prélèvements sur les animaux. Au-delà des questions liées à la recherche,

l'élevage, mais également en ce qui concerne la faune sauvage, puisque le ministère de la transition écologique et solidaire a lancé il y a quelques semaines une grande concertation sur le sujet, et un plan d'action dédié sera effectif dès la rentrée 2019. La parole est Madame la secrétaire d'État, l'élevage français souffre et les éleveurs reçoivent de plein fouet la réaction des Français qui découvrent ces images. La filière viande est excessivement attaquée, notre agriculture est incomprise : nous devons aider le monde agricole à rester digne

Ma question s'adresse à Mme la ministre des outre-mer. Depuis le 3 juin, Mayotte est encore plus isolée qu'à l'ordinaire. L'un des deux 787-8, seuls avions de l'unique compagnie qui assure la liaison directe avec Paris, est immobilisé pour au moins deux mois. Un contrôle a détecté une nouvelle détérioration précoce et inattendue des ailettes du moteur, déjà sous surveillance depuis l'inspection imposée l'an dernier à l'ensemble des opérateurs de ce type d'avion équipé de moteurs Le recours en urgence à l'affrètement d'avions d'autres compagnies est retardé, car il faut assurer aux pilotes une formation sur simulateurs adaptée aux spécificités de la piste courte de Pamandzi. Il en résulte une perturbation des vols, malvenue en cette période estivale.

Tout cela désorganise la vie économique de l'île. Depuis des années, les Mahorais réclament en vain l'aménagement d'une piste longue qui permettrait le désenclavement de l'île.

que Mayotte, ils paient leurs billets d'avion très cher et sont à la merci de tout souci technique, sans solution de rechange. L'apparition brutale d'un volcan sous-marin près de Mayotte avec une menace de submersion ou de tsunami, en premier lieu là même où se trouve l'aéroport, complique encore la donne. Il faudra trouver et mettre en oeuvre sans tarder des solutions innovantes. Dans ce contexte difficile, madame la ministre, quelles actions envisagez-vous ?

Monsieur le Premier ministre, lors de votre discours de politique générale, vous avez une fois de plus appelé l'agriculture française à changer de modèle. Or, à force de critiquer notre modèle ces dernières années et de distiller ce message, vous amplifiez son déclin La production agricole française stagne en volume, alors que celle de nos concurrents augmente. L'excédent commercial agricole a été divisé par deux en cinq ans, et risque de disparaître en 2023.

Un légume et un fruit sur deux sont importés, ainsi qu'un quart du porc. Et même le jambon bio vient d'Espagne ! Monsieur le Premier ministre, êtes-vous conscient de cette réalité ?

Les services régionaux réalisent 5 000 prélèvements par an sur les végétaux placés sur le marché. En 2017, le taux de non-conformité des produits soumis à un contrôle renforcé à l'importation s'élève à 9,3 %. Il est lié soit à la présence de résidus d'un produit non autorisé, soit au dépassement

Les LMR sont calculés pour chaque denrée et chaque substance, afin d'assurer un traitement efficace et une alimentation saine. Comme l'a constaté la DGCCRF, la fraude semble plus importante pour les produits importés issus de l'agriculture biologique, ce qui pose un problème de relation de confiance à l'égard des consommateurs. Le Gouvernement met tout en oeuvre pour lutter contre cette concurrence déloyale

La réalité, monsieur le ministre, c'est que plus vous opposez les modèles, plus vous favorisez l'agribashing, alors qu'un tiers des agriculteurs a plus de 55 ans et qu'il faudrait renouveler les exploitants La réalité, c'est que plus vous contraignez nos agriculteurs sans suffisamment contrôler les importations, plus vous ouvrez la porte à des produits qui ne respectent pas les normes françaises ! La réalité, c'est que changer de modèle et monter en gamme se traduira par une segmentation des Français

que la réalité de son action est faible. Alors, monsieur le ministre, j'en appelle à votre bon sens : arrêtez ce jeu de massacre suicidaire pour notre agriculture française !

qu'il portait déjà sur le déficit de l'assurance chômage et sur les contrats courts- les négociations se sont certes déroulées sous un autre gouvernement, mais dans lequel figurait Emmanuel Macron -, et que vous ne lui avez pas laissé sa chance ? Me confirmez-vous qu'un accord avait été trouvé le 22 février 2018 sous votre mandature, qu'il portait également sur les contrats courts et la gestion de la dette, et que vous avez balayé les propositions des partenaires sociaux ? Me confirmez-vous, enfin, que le scénario alarmiste que vous évoquez, qui serait lié à la dette de l'assurance chômage, n'est pas réaliste et que l'Unédic prévoyait un retour à l'équilibre du dispositif au deuxième semestre 2020

donc dans le strict respect de la loi, madame la sénatrice : la loi prévoit que si les partenaires sociaux ne parviennent pas à définir les règles de l'assurance chômage, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous prenons donc nos responsabilités

samedi dernier, en Savoie, syndicats, associations et partis manifestaient contre l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques. L'injonction de la Commission européenne à privatiser la gestion des barrages dans le cadre du renouvellement des concessions se voit donc opposer une réprobation citoyenne et transpartisane pour défendre à la fois la gestion publique et notre bien commun qu'est l'eau. Un consensus se dessine pour rejeter l'ouverture à la concurrence de ce secteur stratégique d'avenir qui dégage un bénéfice net de 1,25 milliard d'euros par an. Les barrages produisent une énergie vertueuse, décarbonée, garante de notre indépendance et disponible immédiatement. Ils jouent de plus un rôle essentiel dans la compensation des variations de production en apportant une réponse fiable à la perte d'inertie des systèmes. Ils permettent enfin de stocker le surplus d'électricité. Bref, leur rôle est central et indispensable pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Notre pays tire aussi de nombreux avantages qui dépassent le seul intérêt énergétique : irrigation, soutien au débit d'étiage, gestion des crues. Quatre cents barrages, en majorité gérés par EDF, sont concernés par la mise en concurrence. Nous pouvons avoir un doute sur la gestion, qui sera certainement purement comptable, des futurs opérateurs : ainsi, rien ne nous assure que les opérateurs en question continueront à fournir de l'électricité pendant les périodes moins rentables. Peut-on brader au plus offrant un patrimoine vertueux, qui fonctionne, qui est sécurisé et a été financé par les Français ? À la fin, tout est-il marchandise ? Quelle est votre religion sur cette ouverture à la concurrence ?

le Premier ministre l'a dit lors de son discours de politique générale : la France soutiendra son modèle d'hydroélectricité, qui, comme vous l'avez rappelé, est la première source d'énergie renouvelable, afin de garantir les enjeux d'intérêt public lors du renouvellement des concessions. Dès 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu des mesures protectrices pour les salariés des concessions hydroélectriques, à savoir le maintien de leur statut et la reprise à des conditions équivalentes en cas de nouveau concessionnaire.

Le Gouvernement continue de contester l'idée d'une rupture d'égalité sur le marché de la fourniture d'électricité au détail et l'idée d'un quelconque avantage discriminatoire Par ailleurs, je vous rejoins : les barrages hydroélectriques, les concessions hydroélectriques constituent des enjeux sociaux, économiques, écologiques majeurs, liés à l'hydroélectricité, en particulier à la gestion de l'eau et à la sécurité des ouvrages. » ... ... le principe de mise en concurrence des concessions échues découle du droit national et européen. Le Gouvernement s'y prépare en défendant des principes essentiels, notamment en s'opposant à toute interdiction de candidater pour EDF et à la remise en concurrence des concessions non échues. C'est la défense d'une application équilibrée de la loi relative à la transition énergétique : regroupement des concessions dans une même vallée, prolongation de certaines concessions dans le respect du droit, possibilité de constituer des sociétés d'économie mixte lors du renouvellement des concessions, lorsque les collectivités locales sont intéressées. Les échanges avec la Commission européenne se poursuivent, mais aucun accord n'a été trouvé à ce stade. Nous défendrons les intérêts généraux des concessions hydroélectriques dans ce débat. Nous prenons acte de votre réponse et serons particulièrement vigilants sur ce sujet, madame la secrétaire d'État. Je tiens à rappeler que certains de nos voisins n'ont pas de régime concessif et ne seront donc pas concernés par la mise en concurrence. Je tiens également à préciser que le renouvellement des concessions dans certaines vallées pourrait remettre en cause l'équilibre patiemment construit : nos territoires ruraux n'ont pas besoin de cette menace

par heure a été prise sans tenir compte des besoins de nos concitoyens dans leur vie au quotidien et des problèmes spécifiques aux zones rurales. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait provoqué des réactions de colère qui ont été en grande partie à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Tout comme d'autres parlementaires, je me suis opposée à cette mesure impopulaire. La solution que nous avons adoptée au Sénat consiste à assouplir le dispositif en donnant aux préfets et aux présidents de département le pouvoir de rétablir la limitation de vitesse sur les routes nationales et départementales lorsqu'il n'y a pas de danger particulier. Or on s'achemine vers une mesure, qui est incohérente, puisque le seuil des 80 kilomètres par heure resterait obligatoire sur toutes les routes nationales, les routes départementales étant les seules susceptibles de bénéficier d'un retour au seuil des 90 kilomètres par heure. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous justifier une telle discrimination entre routes nationales et routes départementales ? Par ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il serait plus sage et plus cohérent de conserver une norme nationale à 90 kilomètres par heure et de permettre,, aux préfets et aux présidents de département de limiter la vitesse à 80 kilomètres par heure dans les endroits les plus accidentogènes ?

c'est une évidence -toutes leurs responsabilités. et l'inscrire dans le code de la route serait une mesure de bon sens.

le Conseil européen des 20 et 21 juin derniers a permis aux chefs d'État et de gouvernement d'aborder de nombreux sujets. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous avant ce Conseil. Nous avions alors constaté que l'agenda s'annonçait chargé. Les commentateurs Les commentateurs ont volontiers retenu la seule question des nominations, en négligeant parfois les avancées importantes que nous avons enregistrées sur d'autres points, sur lesquels je voudrais revenir. Pour

comme l'a redit le président du Conseil européen, Donald Tusk, à l'issue de la réunion, aucun des trois candidats identifiés par cette procédure - Manfred Weber pour le PPE, Frans Timmermans pour les socialistes et Margrethe Vestager pour le groupe centriste

Ce n'est pas une bataille de drapeaux. Si nous nous plaçons sur le terrain de la bataille d'influence nationale, le projet européen ira dans le mur. Il s'agit avant tout d'une bataille de crédibilité, pour que l'Europe puisse peser et prendre des décisions efficaces au cours des cinq prochaines années.

Les quatre grandes priorités identifiées dans ce programme ont fait l'objet d'un large consensus parmi les États membres : protéger les citoyens et les libertés ; mettre en place une base économique solide et dynamique construire une Europe neutre pour le climat, verte, équitable et sociale ; et promouvoir les intérêts et les valeurs de l'Europe sur la scène mondiale. Ce programme stratégique fixe ainsi un cap clair, qui correspond pleinement aux priorités défendues par la France depuis maintenant plusieurs années,

Sur cette base, les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus d'avoir un nouvel échange de vues sur ce sujet en octobre prochain, dans la perspective de parvenir à un accord avant la fin de l'année 2019.

aux, et améliorer la capacité de réaction de l'Union face aux menaces hybrides et cyber. À la demande de la France, le Conseil a invité les institutions de l'Union européenne, ainsi que les États membres, à oeuvrer à des mesures visant à renforcer la résilience et à améliorer la culture de sécurité de l'Union européenne, notamment pour mieux protéger les réseaux d'information et de communication de l'Union, ainsi que ses processus décisionnels, contre les actes de malveillance de tout type.

en appelant à le développer davantage. Il a également souligné le caractère essentiel pour l'Union de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité des pays de la rive sud de la Méditerranée.

Le Conseil européen a par ailleurs décidé de renouveler, pour six mois supplémentaires, les sanctions sectorielles européennes appliquées à la Russie. Ces dernières sont non pas une fin en soi,

À cet égard, les chefs d'État ou de gouvernement ont salué les progrès réalisés par l'Eurogroupe sur la révision du traité sur le mécanisme européen de stabilité, qui vise notamment à faciliter l'utilisation de ce mécanisme en cas de crise,

une discussion en format article 50 a été organisée à l'issue du Conseil européen pour évoquer la situation du retrait britannique depuis le sommet du 10 avril.

pas ne pas évoquer la défense, au lendemain du salon du Bourget où a été signé l'accord avec l'Allemagne et l'Espagne sur l'avion de combat du futur, et à la veille de l'examen, en commission des affaires étrangères, du traité d'Aix-la-Chapelle.

La réaffirmation symbolique de l'amitié franco-allemande est, nous en sommes tous d'accord, une nécessité absolue dans un contexte marqué par le Brexit et la montée des rivalités entre puissances. Le moment est bien choisi pour donner un successeur au traité de l'Élysée de 1963, car l'amitié franco-allemande est non seulement la grande réussite de l'après-guerre, mais surtout, aujourd'hui, le socle de la pérennité de l'Union européenne. Vous connaissez notre préoccupation sur un volet essentiel du traité : la coopération sur les programmes de défense, clé de l'indépendance stratégique européenne future. Au-delà de la volonté d'avancer manifestée par le texte et les dirigeants des deux côtés du Rhin, de nombreuses incertitudes pèsent sur les projets communs, qu'ils concernent les avions, les drones ou les chars lourds. Je parle évidemment de la politique d'exportation. On ne peut vouloir construire un avion de combat européen ensemble et tout faire pour qu'il soit impossible de l'exporter. C'est une question de cohérence Les bisbilles du partage industriel ne doivent pas empêcher la défense européenne d'avancer. Le Président de la République et la Chancelière l'ont clairement dit, c'est 50-50, et on pourra exporter librement. Tels sont les principes ! Appliquons-les

Oui, nous condamnons l'annexion de la Crimée ; oui, nous demandons l'application des accords de Minsk et la libération des marins ukrainiens ; oui, nous demandons aux Russes de modérer leurs alliés iraniens et d'agir sur leur allié syrien pour mettre fin à l'atrocité des bombardements à Idlib. Cependant, Cependant, la Russie est un grand partenaire stratégique, au coeur de la résolution des crises au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Il est tout de même invraisemblable de constater qu'on parlait davantage aux Russes

ouvrir un nouvel espace de dialogue avec la Russie. La réintégration de la Russie au sein du Conseil de l'Europe, dont le principe a été adopté hier soir, permettra aux citoyens russes opposants

secrétaire d'État, vous avez indiqué la semaine dernière que la question de l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord ne serait finalement discutée qu'en octobre, dans l'attente d'une position du Bundestag. Mais vous n'avez pas clairement exprimé la position que la France adoptera à ce sujet. La Commission européenne met en avant les progrès effectués par ces deux pays. Il nous faut bien sûr éviter qu'ils ne basculent sous d'autres influences- ici même, nous recevons leurs représentants quasiment chaque semaine.

Mais l'Union européenne ne nous semble pas prête à accueillir de nouveaux membres ! Non, ça suffit ! Elle se débat toujours avec le Brexit et avec sa propre refondation. Là est, aujourd'hui, la priorité : refonder l'Europe

Voilà l'Union européenne prête à prendre des sanctions à l'égard d'un État qui est un candidat à l'adhésion depuis plus de trente ans. Nous saluons la fermeté du Conseil face aux activités de forage illégales en Méditerranée orientale et en mer Égée, facteur de déstabilisation pour plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment la Grèce et Chypre, où j'irai moi-même dans quarante-huit heures. Mais la Turquie est un partenaire stratégique, membre de l'OTAN. Notre coopération antiterroriste est essentielle. Nous avons besoin de la Turquie dans la gestion des migrations. Il y a peu de chances de voir les menaces de sanction faire effet- vous l'avez dit vous-même, madame la secrétaire d'État ! Qu'a-t-on à gagner à éloigner chaque jour un peu plus la Turquie de l'Union européenne ? Les dirigeants turcs ne sont pas le peuple turc on le constate au résultat des élections municipales d'Istanbul. Et les électeurs turcs ne sont peut-être pas aussi naïfs qu'on le pense ! Quelle sera donc la position du Gouvernement ?

compliquée que vit et que va vivre l'Europe avec le Brexit, nous devons évidemment adopter, sur tous ces sujets, des positions claires. Le Sénat est prêt à vous accompagner

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la réunion du Conseil européen qui s'est tenue la semaine dernière, la première depuis les élections européennes, était très attendue pour fixer le cap de l'Union européenne jusqu'en 2024. Or, loin de tenir ses promesses, cette réunion a surtout confirmé l'existence de divergences majeures entre les États membres, le Conseil européen renvoyant d'ailleurs à une date ultérieure la prise des décisions concernant les principaux sujets intéressant la commission des finances.

Certes, le temps européen relève du temps long, et le prochain cadre financier pluriannuel déterminera les moyens financiers de l'Union européenne jusqu'en 2027. Toutefois, ce retard pèsera nécessairement sur les conditions de démarrage des programmes nationaux bénéficiant des fonds européens, alors que ceux de l'actuelle programmation ont déjà pâti de difficultés importantes. Espérons, madame la secrétaire d'État, que la présidence finlandaise trouvera une issue favorable à ces négociations. Elle dispose pour cela d'un délai serré. Deuxièmement, à défaut de réussir à s'accorder sur la nomination du futur président de la Commission européenne, et, plus globalement, sur la répartition des nominations aux postes clés des institutions européennes, les vingt-sept États membres ont adopté un programme stratégique pour les années à venir. Ce programme stratégique vise à orienter les travaux des institutions européennes au cours des cinq prochaines années. Il s'articule autour de quatre priorités, dont celle de construire une « base économique solide et dynamique » ; reste à savoir qui l'incarnera. Ce programme sans apporter de propositions concrètes, maintient l'approfondissement de l'union économique et monétaire au rang des priorités de l'Union européenne. Or l'affirmation de cette priorité contraste quelque peu avec les conclusions du sommet de la zone euro qui s'est tenu vendredi en format élargi.

trouvé sur la capacité budgétaire de la zone euro, abandonnant ainsi la fonction de stabilisation de ce budget que préconisait la France depuis deux ans maintenant. Madame la secrétaire d'État, je ne reviendrai pas sur l'ampleur et l'utilité réduites de ce nouvel instrument budgétaire. Le président de la commission des finances, Vincent Éblé, a lui-même, en la matière, exposé ses réserves la semaine dernière. États membres se sont en revanche accordés sur la nécessité de progresser s'agissant du troisième pilier de l'union bancaire, à savoir le système européen de garantie des dépôts. Pour rappel, en décembre 2015, la commission des finances avait déjà adopté une proposition de résolution sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire, dans laquelle elle avait souligné l'effort contributif

Il semble donc peu réaliste de croire à un accord à brève échéance. Enfin, les États membres ont validé l'accord de l'Eurogroupe relatif à la réforme des statuts du mécanisme européen de stabilité, le MES. Ce dernier devrait constituer un filet de sécurité du Fonds de résolution unique d'ici à 2024. La commission des finances a déjà salué les progrès réalisés en ce sens, permettant de renforcer la résilience de notre système bancaire. Toutefois, je veux attirer votre attention, madame la secrétaire d'État, sur le poids des contributions des banques françaises au Fonds de résolution unique. En 2018, celles-ci ont représenté 2,3 milliards d'euros au total.

La montée en puissance du Fonds de résolution unique doit s'accompagner de règles claires du calcul des contributions, afin de rendre le montant de

Comme vous aviez pu le constater lors de notre débat de jeudi dernier, madame la secrétaire d'État, notre commission avait de fortes attentes à l'égard de la réunion du Conseil européen qui s'est tenue les 20 et 21 juin. Sans doute certaines de ces attentes sont-elles déçues à l'issue de ce sommet ; en effet, cette réunion n'aura pas permis de faire émerger les noms des futurs dirigeants des institutions européennes. Il est un peu tôt pour savoir si le Conseil européen a définitivement enterré le processus des, prévu pour consacrer la tête de liste du groupe parlementaire européen sorti le plus puissant des urnes. des urnes. Restent ouvertes à ce jour, en tout cas, certaines options que la France pourrait valablement soutenir. Il est encore possible de nommer, comme nous l'espérons, des personnes expérimentées et crédibles aux postes de président de la Commission, de président du Conseil ou de Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le Gouvernement aurait voulu faire de l'Europe un fer de lance dans cette perspective. Mais le Conseil européen a malheureusement échoué à s'accorder sur l'échéance de 2050 pour parvenir à la neutralité carbone. ailleurs du cadre financier pluriannuel, de l'élargissement ou même du Brexit, les chefs d'État et de gouvernement ont renvoyé ces dossiers au mois d'octobre. Bref, les sujets épineux restent devant nous. Pourtant, le bilan de cette dernière réunion du Conseil européen est loin d'être maigre. L'agenda stratégique de l'Union européenne pour les cinq prochaines années a été arrêté. Il s'organise autour de quatre priorités la protection des citoyens et des libertés, le développement d'une base économique solide pour l'Union européenne, la construction d'une Europe verte, juste et sociale et la promotion des valeurs et des intérêts de l'Europe dans le monde. Il trace une route claire et ambitieuse pour l'Union, qui nous semble adaptée aux immenses défis auxquels celle-ci est confrontée : transition climatique, pression migratoire, extraterritorialité du droit américain, concurrence de la Chine, atteintes au multilatéralisme, menace terroriste, affirmation des mouvements populistes, enjeux de la numérisation. Le Conseil européen n'est en outre pas resté muet sur les tensions internationales du moment, alors que la voix de l'Europe est attendue : il a réaffirmé la primauté des accords de Minsk face aux récentes provocations russes en Ukraine ; il n'a pas passé sous silence les forages menés par la Turquie dans la zone économique exclusive de Chypre- il a ainsi chargé la Commission et le Service européen d'action extérieure de lui proposer des mesures de nature à porter un coup d'arrêt à ces incursions inadmissibles dans le territoire d'un État membre de l'Union. Il a également rappelé l'importance de la politique de voisinage, à l'Est comme au Sud, appelant à se rapprocher des pays de l'autre rive de la Méditerranée, particulièrement le Maroc, mais aussi du continent africain dans son ensemble. Le sommet de la zone euro en configuration élargie qui a suivi la réunion du Conseil européen offre aussi certains motifs de satisfaction : il a entériné la création d'une capacité budgétaire pour la zone euro. Sa voilure est certes réduite par rapport aux ambitions françaises, mais il constitue un premier embryon décisif d'un dispositif que nous appelions de nos voeux depuis longtemps. A également été affirmée la nécessité de poursuivre l'approfondissement de la zone euro dans deux directions la réforme du mécanisme européen de stabilité et l'établissement du fonds européen de garantie des dépôts. Il était important de rappeler ces objectifs pour continuer de consolider la monnaie unique, qui en a besoin.

S'agissant en particulier de la prestigieuse Commission européenne, le système des étant visiblement hors-jeu, et faute de règles très précises dans les traités, seule subsiste la nécessité de parvenir à un consensus le plus large possible entre les membres du Conseil européen, afin que la nouvelle mandature ne s'ouvre pas sur les traces de désaccords. On sait que la désignation du candidat à la présidence de la Commission résulte, d'une part, d'un équilibre au sein de l'ensemble des nominations, et, d'autre part, des souhaits de certains États membres particulièrement proactifs en raison de leur poids politique.

Aussi, sans méconnaître le résultat du PPE, le parti populaire européen, il me semble que le recentrage politique au centre ne doit pas être ignoré, non plus que le renforcement du pôle des écologistes. En attendant, qui que soient ceux ou celles qui seront à la tête des grandes institutions, l'Europe est avant tout un projet à porter. Dans cet esprit, on peut déjà se réjouir que le Conseil européen ait adopté l'agenda stratégique pour les cinq prochaines années. Soucieux de l'approfondissement des politiques communautaires, le RDSE adhère naturellement à la plupart des grandes priorités affichées dans ce cadre. En effet, dans le monde de plus en plus ouvert qui est celui d'aujourd'hui, comment ne pas souscrire aux grandes lignes que la Commission a rappelées à Sibiu en mai dernier : promouvoir les valeurs européennes, protéger les citoyens et les libertés, développer un tissu économique fort et stable et construire une Europe sociale, juste, verte et neutre ? Mais tout cela suppose de surmonter les fractures qui ralentissent, quand elles ne la bloquent pas, l'avancée d'un Nous l'avons d'ailleurs hélas constaté, s'agissant de l'objectif d'une Europe durable, avec la question du climat, qui était un des principaux points à l'ordre du jour de la réunion du Conseil européen. En effet, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à s'entendre. En tout cas, la formule retenue dans les conclusions du Conseil européen est un peu légère : « assurer une transition vers une Union européenne climatiquement neutre ». Que devient, dans ces conditions, l'objectif de neutralité carbone à l'Union européenne, tant dans la perspective du sommet sur le climat prévu en septembre prochain qu'au regard de la mobilisation croissante de la jeunesse européenne sur ce sujet- cet intérêt s'est vraisemblablement manifesté dans les urnes le 26 mai dernier, ne l'oublions pas.

Le Conseil européen s'est également penché sur le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, qui soutiendra notamment l'agenda stratégique. On sait que les négociations sont difficiles, car, là aussi, si les États membres partagent un grand nombre d'objectifs, lorsqu'il s'agit d'entrer dans les détails, chacun avance ses propres priorités. Nous devons reconnaître que la France a les siennes. En effet, est-il utile de rappeler ici, au Sénat, que notre pays est particulièrement attaché au maintien d'une PAC, ou politique

Mais je ne doute pas que le Gouvernement continuera à défendre la PAC et les programmes de cohésion, deux politiques chères au Sénat. S'agissant toujours de la question financière, je m'interroge aussi sur l'articulation du futur instrument de capacité budgétaire de la zone euro, destiné à conforter la compétitivité,

Comme vous le savez, mes chers collègues, l'Union européenne envisage de renforcer sa réglementation en matière de cybersécurité, et le Conseil européen, le 18 octobre dernier, avait préconisé des mesures fortes, dont des mesures restrictives, permettant de décourager les cyberattaques. Où en sommes-nous de ces mesures, des moyens dévolus à l'Agence européenne de la cybersécurité et de la mise en oeuvre d'un système de certification de cybersécurité à l'échelle de l'Union européenne ? ? La sécurité, c'est aussi et bien sûr celle qui doit être assurée à nos frontières et au-delà, les actions que mène l'Union européenne en matière de relations extérieures. Je m'arrêterai sur un seul point : la question des sanctions économiques contre la Russie, que le Conseil européen a décidé de reconduire pour six mois. Il me semble que la reconduction est un bon compromis entre l'assouplissement et le durcissement, compte tenu des incidents en mer d'Azov. Le RDSE est pour sa part attaché à une position d'équilibre permettant de ne pas bloquer la situation sur le plan diplomatique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le Conseil de l'Europe a décidé, cette nuit, de rouvrir ses portes à la Russie. Du côté ukrainien, la présidence Zelensky va-t-elle ouvrir une nouvelle ère et relancer l'application des accords de Minsk, sachant que les relations avec la Russie sont compliquées ?

d'État, mes chers collègues, je veux profiter de cette intervention pour regretter que la France cautionne une politique très partisane de l'Europe,

Le 18 juin dernier, le conseil des affaires générales, à la réunion duquel vous participiez, madame la secrétaire d'État, a « pris bonne note de la recommandation de la Commission d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la République de Macédoine du Nord et l'Albanie, compte tenu de son évaluation positive des progrès accomplis ». Ces conclusions ont été reprises par le Conseil européen, dont la réunion qui s'est tenue le lendemain fait l'objet du présent débat. Je me réjouis vivement de ces déclarations, même si je regrette que nous devions encore attendre le Bundestag pour que le Conseil puisse se prononcer véritablement sur le fond. L'élargissement rapide de l'Union vers les Balkans occidentaux est en effet une évidence historique et culturelle. Lors des conférences que j'ai données en septembre 2018 en Albanie, à Tirana et à Korça, et en Macédoine du Nord, à Skopje, la question : quelle différence y a-t-il entre un Albanais ou un Macédonien du Nord et un Français ou un Allemand ? Aucune : ils sont tous européens deux pays de nous rejoindre est une nécessité stratégique, tant pour l'Union européenne que pour lesdits pays. Ils ne rêvent que d'Europe. Leur fermer la porte serait les inviter à construire leur avenir avec des pays qui combattent notre projet et nos valeurs, comme la Russie, n'en déplaise à M. Masson, la Chine ou la Turquie.

Elle y est même parfois incitée- ainsi les médecins albanais sont-ils systématiquement encouragés à apprendre l'allemand pour exercer chez notre voisin.

L'ancien président a formulé le souhait que nos deux pays tissent des liens plus étroits et que la France accorde davantage d'importance à la région des Balkans. Il craint que notre absence n'offre un espace à d'autres pays. Je lui ai fait part de ma crainte que la jeunesse de son pays ne quitte l'Albanie, au cas où celle-ci ne rejoindrait pas à court terme l'Union européenne. Beaucoup de responsables politiques des Balkans occidentaux partagent cette préoccupation. L'ancien président m'a rappelé que l'adhésion à l'Union européenne est au coeur des aspirations du peuple albanais et, plus particulièrement, de la jeune génération. Ce parcours d'adhésion est jalonné de nombreux défis. L'Albanie consent déjà à beaucoup d'efforts pour y parvenir, à l'image de la lutte contre la corruption, objet d'une réforme de son système judiciaire. J'ai salué ce volontarisme et assuré l'ancien président de mon total soutien à la démarche d'adhésion à l'Union européenne de son pays. évoquer et saluer les efforts du peuple de Macédoine du Nord, qui a accepté de modifier le nom de son pays, par référendum, pour pouvoir accéder à l'Union européenne. Il est temps désormais pour l'Union d'adopter une position claire envers ces pays et envers ces peuples. Madame la secrétaire d'État, la France va-t-elle accepter d'ouvrir des négociations d'adhésion

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous le savions, ce sommet européen était principalement dédié à la distribution des hauts postes institutionnels ; pourtant, malgré de longues discussions, aucun consensus n'a pu être dégagé entre les États membres. Cela n'est pas vraiment une surprise, tant les négociations sur ce sujet sont délicates et l'équilibre difficile à trouver. Nous l'avions souligné lors de notre débat préalable : cette réunion du Conseil européen devait être un moment fort de la démocratie européenne, l'occasion d'affirmer le rôle politique politique de l'Union européenne. Partie remise, donc, au sommet de crise du 30 juin, deux jours seulement avant la session inaugurale du Parlement européen- troisième sommet depuis les élections européennes, des tentatives de compromis, il semble bien que le système du, si critiqué par certains, soit définitivement mort. Les favoris pour la présidence de la Commission ont été écartés, faute d'une majorité parmi les dirigeants de l'Union européenne. Le fait que les chefs d'État et de gouvernement ne se soient pas mis d'accord peut être considéré comme un échec. Cela peut aussi être interprété comme le signe d'une volonté politique de trouver les personnalités adéquates pour diriger l'Union européenne, des femmes et des hommes politiques forts qui feront consensus et qui mettront en oeuvre les priorités définies, répondant aux attentes des citoyens. Il faut des personnalités qui ont déjà exercé des fonctions à responsabilité au plus haut niveau. Je ne peux, à ce titre, que soutenir le Président de la République face à la chancelière allemande, qui veut imposer M. Weber. À la tête de la Commission européenne, il faudrait une personnalité forte qui fasse l'unanimité et qui soit connue du grand public. Et pourquoi pas une femme Il faudra aussi que le président ou la présidente de la Commission européenne s'entoure d'une équipe solide, compétente et approuvée dans son ensemble par le Parlement européen pour mettre en oeuvre les nombreuses priorités européennes. En ce sens, l'agenda stratégique qui a été adopté pour les cinq prochaines années par le Conseil européen guidera la prochaine Commission européenne. C'est écrit noir sur blanc : il faudra protéger davantage les citoyens, développer le tissu économique, construire une Europe sociale, juste et verte, et renforcer les intérêts européens à l'échelon mondial. Autant de dossiers qui mériteront une attention particulière des institutions européennes Le climat en fait partie. Et même si les Vingt-Huit n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la date de 2050 pour la neutralité carbone européenne, les progrès réalisés par la France pour convaincre de nombreux États membres peuvent être soulignés. Il est aussi important de comprendre les raisons du refus de certains États pour adopter une stratégie ambitieuse qui sera acceptée par tous. La Finlande, qui tiendra bientôt les rênes de la présidence tournante de l'Union européenne, a récemment annoncé qu'elle visait des émissions nettes zéro d'ici à 2035 et voulait devenir un pays à bilan carbone négatif d'ici à 2050. C'est encourageant. Madame la secrétaire d'État, le message porté par l'Europe au sommet des Nations unies en septembre prochain devra être fort et audible pour que les signataires de l'accord de Paris renforcent leur ambition en matière de climat. L'approfondissement de l'Union économique et monétaire sera également essentiel dans les années à venir. Les premières pierres posées lors du sommet de la zone euro sont autant de signes encourageants, même si tout n'est pas encore réglé. La question du financement est, certes, compliquée, mais essentielle si l'Union européenne veut avancer concrètement sur cet instrument budgétaire pour la compétitivité et la convergence. C'est en tout cas un pas important qui est franchi pour le budget de la zone euro. Cela devrait permettre d'encourager les réformes structurelles pour accroître la compétitivité des dix-neuf États membres ayant adopté la monnaie unique. Il faudra poursuivre ces travaux pour définir clairement l'architecture du futur budget de la zone euro. Madame la secrétaire d'État, le sommet du 30 juin sera fondamental pour l'avenir de l'Union européenne. Je suis certaine que la France se montrera à la hauteur des enjeux. Gageons que les chefs d'État et de gouvernement réussiront à se mettre d'accord au-delà de leurs intérêts nationaux pour préserver et renforcer notre Europe. La parole

à cette rencontre, les chefs d'États et de gouvernement ont formellement adopté l'accord sur la création d'un budget de la zone euro conclu le 14 juin par les ministres des finances de la zone euro. Cet accord, dont notre groupe se félicite, est une bonne nouvelle. Il marque un pas de plus vers le renforcement des investissements et de la convergence entre les dix-neuf économies de la zone euro, pour leur permettre de mieux résister aux chocs économiques. En effet, l'accord vise trois mesures majeures. D'abord, pour la première fois, un budget opérationnel sera mis en place, afin d'encourager des réformes favorisant la convergence entre économies. Ensuite, le renforcement du Mécanisme européen de stabilité le transformera en un véritable pare-feu d'intervention rapide et efficace en cas de crise. Enfin, la création d'un filet de sécurité en cas de crise est une nouvelle forme de protection des économies des épargnants français, comme de ceux de toute la zone euro. C'est un engagement du Président de la République, énoncé dans son discours de la Sorbonne. Comme il l'a évoqué à la sortie du Conseil européen, nous allons « dans la bonne direction », mais il faudra « aller beaucoup

Deuxièmement, le sommet a permis des échanges sur un nouvel agenda stratégique pour les cinq années à venir. Comme vous venez de le rappeler, cet agenda a été adopté à l'unanimité. Il s'inscrit dans la continuité des résultats du sommet de Sibiu du 9 mai et est destiné à orienter les travaux des institutions, au lendemain d'élections européennes déterminantes, alors que le renouvellement des institutions est encore en cours. Les citoyens européens, qui se sont exprimés dans les vingt-huit pays de l'Union européenne, ont notamment voulu attirer l'attention de leurs dirigeants sur la transformation de nos économies et ses conséquences sur leur vie, sur la protection de leurs libertés et des frontières extérieures, ainsi que sur l'urgence climatique. Nous nous réjouissons que cet agenda stratégique ait su prendre en compte à la fois ces attentes fortes et les défis qui s'imposent désormais à l'Europe, en traçant quatre axes prioritaires : la protection des citoyens et des libertés une Europe économiquement solide et dynamique, en passant notamment par une approche plus intégrée autour de la politique industrielle, de la transformation numérique et d'une fiscalité juste et efficace une Europe neutre pour le climat, équitable et sociale ; enfin, la défense des intérêts et des valeurs européennes sur la scène internationale et l'affirmation de l'Europe comme un rempart face aux défis mondiaux. Notre groupe restera bien évidemment vigilant quant à la mise en oeuvre de cet agenda durant les cinq années à venir. Madame la secrétaire d'État, sur ces quatre axes, des dossiers prioritaires vont-ils émerger ? ? Troisièmement, l'un des enseignements cardinaux de ces dernières élections est l'affirmation saine et massive de la préoccupation environnementale. Celle-ci ne s'est pas seulement exprimée en nombre de sièges. Elle s'est aussi durablement installée au coeur du débat pour chacune des formations politiques en jeu. Et elle continuera de s'exprimer ainsi, à la manière d'une force bienveillante ... et pas souvent tranquille Les revendications pleines d'espoir de notre jeunesse en attestent. Notre groupe se réjouit que le Conseil européen ait su faire écho à une telle préoccupation en inscrivant ce sujet brûlant à son ordre du jour et en adoptant des conclusions spécifiques. Ces conclusions invitent le Conseil et la Commission à faire avancer leurs travaux sur les mesures incitatives et sur le cadre qui permettra d'assurer une transition vers une Union européenne neutre pour le climat, conformément à l'accord de Paris. De même, comme je viens de le souligner, la construction d'une Europe neutre pour le climat, verte et équitable figure bien dans l'agenda stratégique. La France a réussi à franchir une étape supplémentaire, en rassemblant désormais vingt-quatre pays européens autour de l'objectif d'une économie décarbonée pour 2050, pour appliquer pleinement l'accord de Paris. Certains préféreront peut-être voir le verre à moitié vide ; je préfère le voir à moitié plein.

L'espoir nous est d'autant plus permis que, rappelons-le, au sommet de Sibiu, seuls huit pays, et non vingt-quatre comme aujourd'hui, étaient convaincus par l'objectif d'une économie décarbonée d'ici à 2050. Madame la secrétaire d'État, comment réussir à convaincre nos partenaires que sont la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie du bien-fondé d'un tel objectif politique pour nos générations futures ? Surtout quand, nous le savons, les énergies fossiles sont au fondement de leurs systèmes économiques ? Pourriez-vous d'ores et déjà nous informer sur la manière dont la présidence finlandaise compte se saisir de ce dossier ? L'urgence climatique est de mise, et la paralysie politique n'est plus permise. Ce serait la pire des stratégies que d'agir isolément sur ce phénomène global, dans l'attente d'être vertueusement imité. Nous devons donc mettre les bouchées doubles dans les efforts diplomatiques que nous déployons aujourd'hui à tous les niveaux, et demain au G20 d'Osaka des 28 et 29 juin, puis le 23 septembre lors du sommet onusien sur le climat. Il est de notre devoir de combattre la résignation en tout temps et en tout lieu, car le réchauffement climatique, nous nous en rendons bien compte, c'est le déplacement des populations, c'est la guerre de l'eau, c'est aussi l'effondrement de la biodiversité, du monde animal et végétal tel que nous l'avons toujours connu. Madame la secrétaire d'État, quel bilan dressez-vous des efforts diplomatiques multipliés de la France quant au respect et à la mise en oeuvre de l'accord de Paris ? Au Sénat, c'est avec cette conscience que nous prendrons bientôt notre part lors de l'examen du projet de loi relatif à l'énergie et au climat. Nous tenterons de répondre au mieux aux attentes qui se sont exprimées- je pense au poids de l'écologie -lors de ce récent vote.

aussi pour l'avenir des peuples d'Europe, qui attendent des changements importants. Alors que les inquiétants résultats des élections européennes appellent des remises en cause profondes, alors que les revendications sociales, écologiques et démocratiques infusent à travers le continent, tout démarre comme si rien n'allait changer. L'échec du sommet est une alarme de plus sur la crise très profonde de l'actuelle construction de l'Union européenne. Au-delà de la personnalité des candidats aux nominations, au-delà des circonstances, le modèle institutionnel et économique de l'Union européenne est à bout de souffle. Les extrêmes droites de tous poils, dont plus personne ne parle, semble-t-il, exploitent ces impasses répétées pour pousser leurs pions vers une Europe de plus en plus brutale, guerrière, rejetant les solidarités sociales et humaines. Et les chefs d'État conservateurs, néo-libéraux ou sociaux libéraux, incapables de renouveler en profondeur les logiques de l'Union européenne, bloqués dans des institutions et des traités qu'ils ont eux-mêmes façonnés, se révèlent de plus en plus inaptes à résoudre les contradictions et à avancer vers des solutions novatrices. Il y a bien les grandes envolées présidentielles à l'Acropole, à la Sorbonne, devant l'Organisation internationale du travail ou encore au sommet des Deux Rives, mais les réalités sont têtues. Et la réalité, c'est une Europe qui s'enfonce dans la crise, sans projet novateur et sans écoute des demandes citoyennes. Sur les discussions institutionnelles, les mots de Visconti résonnent encore malheureusement : « Il faut que tout change pour que rien ne change. » Le Président de la République se présente comme le pourfendeur des habituelles tractations entre socialistes et conservateurs européens, mais les acteurs restent les mêmes ; seuls les rôles changent. Et pour quel résultat prévisible ? Un nouveau compromis, associant peut-être cette fois un peu plus de libéraux et de verts, mais fondé sur la continuité des mêmes objectifs. Aucun changement de cap sérieux en faveur du progrès social, de la protection de la planète ou d'une nouvelle industrialisation intégrant ces réorientations ! Les arrangements de couloirs reprennent de plus belle sans contrôle des objectifs, loin du regard des citoyens et des parlementaires nationaux. Et, même dans ces conditions, vous n'arrivez pas à déboucher sur un consensus ! La même logique prévaut pour les discussions relatives au cadre financier pluriannuel. Avec le même résultat : un ajournement des décisions. Quels compromis se nouent en arrière-plan des nominations négociées ? Nous voulons de la transparence, une autre méthode et un réel changement de cap. Pourquoi, par exemple, ne pas simplement fonder les priorités budgétaires sur des demandes qui continuent d'être largement exprimées par la grande majorité des citoyens des États membres ? Dans un récent eurobaromètre, la Commission souligne elle-même que la préoccupation première des Européens est celle du développement économique et social, loin devant le développement de la défense européenne. Pourquoi dès lors s'évertuer à faire du fonds européen de défense de 13 milliards d'euros la priorité absolue, sur l'autel de laquelle beaucoup de renoncements à d'ambitieuses politiques sociales semblent se tramer ?

une baisse des montants serait inacceptable, surtout quand on prétend engager le continent dans la transition de nos modèles de production, qui sera impossible sans des revenus redevenus rémunérateurs Une réforme de ces aides est possible et même souhaitable. Il faut limiter les aides versées aux plus grands propriétaires terriens et à l'agriculture la plus productiviste, au profit de modèles de qualité sociale, alimentaire et écologique nouveaux. Mais la mise en cause du montant des crédits de paiements est un véritable danger. La politique de cohésion et, notamment, les divers fonds de solidarité doivent également être sanctuarisés, voire développés vers de nouveaux objectifs de réduction des inégalités. la politique de cohésion est menacée par le projet de cadre financier pluriannuel. Oui, le minimum- je dis bien « le minimum » -serait de protéger les rares dépenses de redistribution qui existent dans l'Union

GUE/NGL, au Parlement européen. Le programme stratégique pour la période 2019-2024 nous alarme, tant il est en décalage avec les grandes urgences de changements nécessaires. Le premier paragraphe est relatif à la protection des citoyens et des libertés ? Très bien Mais quelle est la première idée mise en avant dans ce cadre ? Le renvoi des réfugiés dans les pays d'origine ! Est-ce cela la vision que nous promettons au monde et aux peuples d'Europe à l'aube du XXI siècle ? Et les axes directifs réitèrent tous ceux qui ont clairement échoué. Le Conseil européen appelle à développer notre base économique ? Parfait, il serait temps ! Il mentionne même la politique industrielle. C'est une nouveauté. Mais quel est le principe directeur choisi ? L'investissement public dans des projets utiles ? Des coopérations scientifiques ? Le développement d'une base productive écologique ? Absolument pas !

! Madame la secrétaire d'État, vous l'aurez compris, mon intervention est celle d'un sénateur inquiet pour l'avenir de son continent et des peuples qui le composent. L'installation d'une nouvelle législature est souvent un moment décisif pour engager le changement.

Je crois que le Brexit montre les limites d'une telle méthode. Car, même si nous constatons que nous avons intérêt à ne pas nous séparer, même si nous sommes si interdépendants que nous aurions tous du mal à le faire, nous allons probablement le faire ! Si les le faire ! Si les liens d'interdépendance et les solidarités qui ont été créés ne s'accompagnent pas d'un supplément d'âme qui donne la volonté et la joie d'être ensemble, le danger de la séparation de la déconstruction arrive petit à petit. Ce que nous vivons avec le Brexit est aussi un enjeu majeur pour l'ensemble de la construction européenne à l'avenir. Pourtant, au regard de ce que nous attendions et de ce que les commentateurs annonçaient, le résultat des élections européennes a déjoué les pronostics les plus pessimistes. D'abord, la participation a été plus importante et plus marquante que prévu. Cela montre l'importance que les citoyens accordent à la construction européenne.

le PSE et le PPE n'auront plus de majorité ensemble. C'est aussi un moyen pour que le Parlement européen soit un peu moins dominé par les accords conclus au sein du Conseil européen. Ce sont de bonnes nouvelles. Cela invite à travailler à la démocratisation de l'Europe, qui est la condition de sa future stabilité.

en refusant l'idée que le Parlement européen puisse, par une majorité, choisir le président de la Commission européenne, la France est revenue sur l'acquis démocratique mis en oeuvre en 2014, qui avait permis à une majorité du Parlement européen de choisir le président de la Commission européenne. le Président de la République refuse de reconnaître le rôle et la responsabilité des partis politiques dans la vie démocratique. À Paris comme à Bruxelles, cette attitude représente un risque.

et la neutralité carbone. On ne trouve rien sur la manière dont cette exemplarité sera utile pour faire évoluer l'ensemble de nos partenaires commerciaux. Nous sommes la première puissance commerciale du monde. Nous avons une responsabilité particulière pour que l'ensemble du commerce prenne la voie d'une neutralité en carbone, sans repli sur soi, mais, au contraire,

vertueux. Il faut y travailler avec nos partenaires commerciaux. Rien non plus sur la défense du droit d'asile, qui est le fruit de notre histoire et des promesses de nos anciens : ne jamais revoir les horreurs que nous avons vécues sur le continent. d'un engagement pour une Europe humaniste, combattant pour la liberté. Dans ce projet stratégique, il n'y a rien ! Pourtant, nous le savons, la question du droit d'asile est au coeur des négociations entre les États européens aujourd'hui. Il y a une inquiétude sur l'idée que l'Union se fait de son rôle à ses propres frontières. Nous ne pourrons jamais progresser dans l'approfondissement politique de l'Union européenne si nous laissons des parties entières de nous-mêmes au-delà de nos frontières. Je pense en particulier à la Macédoine, qui a fait, avec la Grèce, de gros efforts ces derniers mois ; ils devraient être salués. Pourtant, le conseil des ministres des affaires étrangères n'a pas mis à l'ordre du jour du Conseil européen l'ouverture des négociations avec la Macédoine. Au lieu d'un budget de la zone euro, on se contente d'une petite ligne de crédit dans un projet de cadre financier pluriannuel, qui n'a pas avancé au cours des négociations. Rien sur l'enjeu du vieillissement de la population, qui pèsera sur notre croissance, mais aussi sur notre capacité d'innovation et sur notre capacité de remettre en cause nos habitudes face aux exigences climatiques. Rien sur l'amélioration des ressources propres de l'Union européenne, alors que le prochain cadre financier pluriannuel est difficile à mettre en place. En effet, chaque cadre financier pluriannuel fait justement de plus en plus appel aux ressources des États plutôt qu'aux ressources propres. Il conviendrait de modifier une telle évolution. Rien Rien sur la manière dont l'Europe, première puissance commerciale du monde, pourrait envisager de faire face à l'extraterritorialité des lois américaines, qui viole notre souveraineté, le droit international et qui menace aujourd'hui aussi la paix. Rien de bien concret sur l'évolution de la politique de concurrence qu'il convient de mettre en place pour répondre aux problèmes que nous avons constatés lors du projet de fusion Alstom-Siemens, alors que la Commission n'a fait que dire le droit.

général sur la protection des données, ou RGPD ; c'est une condition absolument essentielle de notre liberté pour demain. L'Europe, c'est la chance pour les Européens de ne pas se chamailler, de ne pas être des spectateurs de l'évolution du monde, mais d'être ensemble Nous avons aujourd'hui la force, notamment commerciale, de pouvoir faire la norme et de peser sur l'ensemble du monde. Les États membres, au lieu de continuer à défendre les intérêts nationaux, devraient être à la hauteur de ce que les citoyens européens

ainsi que les postures de leurs chefs d'État et de gouvernement. Cela nous inquiète pour l'avenir de la construction européenne. Nous ne pouvons pas faire la démocratisation de l'Europe sans les partis politiques. Nous ne pouvons pas avancer sans respecter une majorité au Parlement européen. Nous ne pourrons pas faire en sorte que cette démocratisation se fasse, si la Commission continue à être un autre club, comme le Conseil européen, réunissant des représentants des États. Non ! La Commission doit être solidairement responsable, choisie par son président, validée par une majorité au Parlement européen et porteuse d'une politique qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui sera le choix de le choix de la majorité des Européens. Très bien dit ! Ce sera beaucoup plus difficile que les fois précédentes, parce que les majorités au Parlement européen seront plus compliquées. Mais c'est aussi pour cela que la démocratisation de l'Europe est possible aujourd'hui, lors de cette législature. Il est de notre responsabilité de la réussir. Pour cela, il faut que les différents gouvernements soient à la hauteur des attentes

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil européen a adopté des conclusions dans plusieurs domaines stratégiques, dont le changement climatique. La hausse des températures est une réalité éprouvée concrètement cette semaine, y compris dans cet hémicycle ! Quelle que soit la température ressentie en ce moment, il est utile d'évoquer, parmi les intérêts stratégiques de l'Union européenne à protéger, le climat. L'Union a tout intérêt à construire une Europe du climat qui ne soit pas en opposition avec le développement économique. Le Conseil européen du 20 juin 2019 affirme que « l'Europe doit s'appuyer sur une approche inclusive et durable, qui tire parti des changements induits par la transition énergétique Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle, à l'origine de bien des politiques européennes. Plus loin, le Conseil européen explique que l'Union doit montrer la voie pour une neutralité climatique en tenant compte des situations nationales tout en étant socialement juste. la quadrature du cercle. Au-delà d'un appel à se conformer à l'accord de Paris, il n'y a rien de concret dans cette feuille de route. Pourtant, nous répétons depuis de nombreuses années que la planète ne peut plus attendre. Le marché européen de l'énergie intégré n'existe pas encore, tant s'en faut. L'accélération de la transition vers les énergies renouvelables est complexe, notamment en France. Par exemple, en 2018, la ferme d'éoliennes offshore la plus puissante du monde a été inaugurée en mer d'Irlande. Il existe plus de 4 000 éoliennes maritimes en Europe, essentiellement réparties au large du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Suède. Il n'y en a aucune sur les côtes françaises.

Je rappelle que le premier appel d'offres pour développer la filière remonte à 2011. Aujourd'hui, ailleurs en Europe, il faut quatre ou cinq ans pour créer un parc éolien en mer. La France double la mise avec des périodes de recours de trois ou de quatre ans supplémentaires. Une telle situation n'existe nulle part ailleurs en Europe. Oui, l'économie circulaire devra s'appuyer sur des partenariats public-privé. Mais une fois qu'on l'a dit et répété, que fait-on ? Quels sont les investissements européens prévus pour les mobilités de demain ? Les conclusions du Conseil européen rappellent aussi la nécessité de préserver les systèmes environnementaux, notamment les océans. Le 2 avril dernier, lors du dernier débat post-Conseil européen, je soulignais que la mondialisation des échanges s'effectuait par les océans, sur des autoroutes maritimes aux équilibres biologiques fragiles, d'où l'importance d'un « espace européen de sécurité maritime » contenu dans le paquet«Erika III ». La création de l'Agence européenne pour la sécurité maritime en 2002 a été utile, mais nous devons améliorer les dispositifs. N'oublions jamais que la souveraineté alimentaire se trouve aussi sur la mer et dans la mer. La préservation des océans est un formidable gisement économique. Je pense, par exemple, aux larges possibilités offertes par les macro-algues et micro-algues alimentaires. Ce sont des aliments naturels produits de manière durable grâce à des procédés innovants. raison de la croissance de la population mondiale, nous devons chercher de nouvelles sources protéiques pour nous alimenter. La mer en regorge. La demande alimentaire mondiale augmentera probablement de 50 % d'ici à 2050. C'est donc une question de sécurité alimentaire. Nous devons également tenir compte de l'augmentation des températures, qui est susceptible de modifier l'équilibre des flores marines. L'enjeu n'est pas mince. Les études du Centre d'études stratégiques de la marine apportent un éclairage utile sur la question de la préservation des océans et des problématiques alimentaires. L'interdépendance entre protection du milieu marin, commerce et sécurité alimentaire est forte. L'Union devrait être un moteur sur cette question éminemment maritime et européenne.

butoir. Le charbon a encore de beaux jours devant lui ! Comment l'Union européenne accompagnera-t-elle la transition énergétique des pays membres les moins riches ? Quels seront les mécanismes de compensation ?

le 21 juin dernier s'est tenu un sommet de la zone euro au cours duquel a été examinée la situation économique de la zone. Il y a notamment été débattu de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Parmi les avancées obtenues ou espérées, j'en retiendrai deux. Tout d'abord, je retiens la mise en place d'un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro. Si celui-ci représente une piste pertinente pour relancer l'activité économique en stimulant l'investissement public, il semble bien éloigné d'un véritable budget de la zone euro tel qu'esquissé lors du discours de la Sorbonne. Un tel outil est pourtant indispensable pour corriger les conséquences des chocs asymétriques et des structures hétérogènes des économies nationales, tout en accompagnant la disparition des politiques monétaires nationales d'une politique budgétaire commune. Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous présenter les ambitions d'un tel « instrument budgétaire » et nous préciser ses sources de financement dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel ? Je retiens ensuite le renforcement de l'union bancaire. Sa mise en place doit nous permettre de protéger les contribuables et les épargnants d'éventuelles défaillances du secteur financier, tout en démontrant qu'un partage de compétences entre États européens peut apporter aux citoyens davantage de protection et de sécurité que l'action isolée d'un État. Toutefois, quelles ont été, madame la secrétaire d'État, les avancées concernant le troisième pilier de cette union, à savoir un système européen de garantie des dépôts ? Sans celui-ci, l'union bancaire aura bien du mal à assurer la stabilité du secteur bancaire. Par ailleurs, le dernier Conseil européen fut l'occasion d'évoquer le nouveau programme stratégique 2019-2024 et d'insister sur la nécessité de concevoir une « politique industrielle permettant d'affronter l'avenir Or je constate que nous sommes pour le moment incapables de passer de politiques industrielles nationales cloisonnées à une politique industrielle européenne à même de faire émerger des géants industriels européens. Pour cette question comme pour tant d'autres, l'Union européenne ne pourra traiter d'égale à égale avec les autres puissances en adoptant une approche morcelée. parvenir qu'en formant un front uni et « en s'appuyant sur ses propres ressources et sur celles des États membres ». Cette question a-t-elle été évoquée, madame la secrétaire d'État ? En outre, ce sujet ne peut que m'amener à aborder celui de la politique européenne de concurrence dont l'obsolescence est dénoncée de tous bords, alors que l'actuelle commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, faisait partie des candidats malheureux à la présidence de la Commission européenne les 20 et 21 juin derniers. Des pistes ont-elles été évoquées pour enfin refonder les règles de concurrence, particulièrement en matière de contrôle des concentrations et d'interdiction absolue des aides publiques, penser une stratégie industrielle européenne intégrée et pour promouvoir des règles du jeu équitables avec les autres grandes puissances, notamment concernant l'application du principe de réciprocité dans les échanges internationaux Enfin, je m'étonne que la plus ancienne et la plus importante des politiques en termes de budget n'ait pas été évoquée lors de ce Conseil européen, alors même qu'elle est à la croisée des enjeux en termes de développement durable, de développement rural et de sécurité. Je parle, bien évidemment, de la politique agricole commune et de sa réforme prochaine. Vous l'avez récemment dit, madame la secrétaire d'État, le premier défi à relever est celui d'une PAC qui protège ses agriculteurs. Le deuxième défi est celui d'une PAC qui protège ses consommateurs. Enfin, le dernier défi est celui de sa simplification. Toutefois, la nouvelle réforme à venir pour la PAC après 2020 en réduit substantiellement le budget tandis que, dans le même temps, elle prévoit également de donner davantage d'autonomie aux États membres. Qu'en est-il, madame la secrétaire d'État, des discussions autour de cette réforme et de ses ambitions pour les prochaines années ? La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil européen s'est accordé sur un programme stratégique pour la période 2019-2024 sur la base de quatre priorités.

à promouvoir les intérêts et les valeurs de l'Europe sur la scène mondiale. Voyons son application pratique dans les relations avec la Russie. Le Conseil européen vient de décider unanimement de renouveler pour une période de six mois les sanctions économiques contre la Russie. Si cette décision n'a rien d'étonnant, il n'en est pas de même de l'absence d'invitation aux cérémonies du 6 juin dernier du président Poutine. L'Allemagne à l'origine de la guerre était invitée, mais pas la Russie, qui a détruit 80 % des divisions du III Reich et sacrifié 27 millions d'habitants pour lutter contre le nazisme. Ce n'est certainement pas un hasard si la réponse du président Poutine à ce camouflet a été de recevoir, ce même 6 juin, dernier le président de la Chine pour renforcer une coopération bilatérale, déjà très étroite. Dans cet état d'esprit, a été annoncé le choix très probable de la technologie chinoise Huawei pour équiper les futurs réseaux 5G en Russie. Le lendemain, le 7 juin, le monde entier a pu découvrir que la flotte russe croisait en mer de Chine aux côtés de la flotte chinoise. d'une quasi-collision entre un navire de guerre russe et un navire de la septième flotte des États-Unis, dont la mission est d'empêcher la Chine de s'approprier les eaux de la mer de Chine méridionale. Il faut tout de même noter que les pays européens qui veulent durcir et prolonger indéfiniment les sanctions contre la Russie, quitte à la pousser ainsi dans les bras de la Chine, sont ceux qui contribuent le moins à la construction de l'Europe de la défense, chère à Emmanuel Macron. La Pologne, la Lituanie et la Lettonie apportent régulièrement par milliards leur contribution au complexe militaro-industriel américain. Aucun pays de l'Union européenne n'a d'ailleurs acheté de Rafale Par ailleurs, les sanctions économiques occidentales ont amené la Russie à rechercher et à atteindre ses objectifs d'autosuffisance alimentaire. En 2017, la Russie est devenue le cinquième exportateur mondial de céréales. Pendant ce temps, les sanctions font perdre aux pays de l'Union européenne près de 5,9 milliards de dollars d'exportations dans le secteur agroalimentaire. Eh oui ! Il est donc temps de faire le bilan diplomatique et économique de la reconduction rituelle des sanctions qui éloignent la Russie de l'Europe au plus grand bénéfice de la Chine. Il est urgent de faire bouger les lignes ! Très bien ! La visite du Premier ministre russe, hier, au Havre, en compagnie de notre Premier ministre, indique qu'Emmanuel Macron s'y emploie. Il a opportunément déclaré au début du mois de juin que « l'Europe a besoin d'une nouvelle grammaire de confiance et de sécurité avec la Russie qui ne doit pas passer exclusivement par l'OTAN ». Alors que la Russie avait menacé de quitter le Conseil de l'Europe, la France a pris en main avec succès la manoeuvre diplomatique pour que la Russie retrouve toute sa place au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le président Macron a également reçu il y a quelques jours le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dont la priorité absolue est le retour à la paix dans l'est de l'Ukraine. Cela suppose la relance du processus de Minsk, que supervisent la France et l'Allemagne,

L'ambition du président Macron de faire enfin jouer à l'Union européenne ou, à défaut, à la France et à l'Allemagne un rôle géopolitique autonome est donc à saluer et à encourager ! La parole est à M. Benoît

au lendemain de ce grand rendez-vous démocratique qu'ont été les élections européennes, et juste après l'adoption lors du Conseil européen des 20 et 21 juin du nouveau programme stratégique, j'interviens dans le cadre de ce débat au Sénat pour dire ma satisfaction, exprimer mes attentes sur l'Union européenne et réaffirmer mes convictions quant à une Union européenne mieux coordonnée et qui s'impose dans un contexte mondial tant déstabilisé. Rarement l'humanité aura eu à faire face à autant de dangers et de défis Nous sommes nombreux à nous réjouir des ambitions européennes, alors que certains dirigeants de grands pays, plus ou moins ouvertement, voulaient détruire la construction européenne et que la machine à fabriquer des était à la manoeuvre pour que l'Union sorte affaiblie de ces élections et marque le pas. C'est finalement l'inverse qui s'est produit. La participation des électeurs a été importante, avec un beau pourcentage de jeunes, et le vote populiste a été contenu. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, tout cela nous engage et nous oblige à ne plus perdre de temps. Si les Vingt-Sept ont été trop accaparés par le Brexit, ils sont néanmoins sortis unis de l'épreuve.

Le plan stratégique adopté la semaine dernière va dans le bon sens en nous donnant les moyens de nos ambitions. Une augmentation et une plus grande mutualisation de nos moyens et de nos savoir-faire permettront de renforcer la performance de tous les secteurs de production industrielle, agricole, alimentaire et de services, y compris dans les domaines de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle. nous permettra d'être un acteur déterminant dans la lutte contre le réchauffement climatique et en faveur du développement durable que nous devons à nos enfants. Dans ce domaine, efforçons-nous cependant d'adopter une démarche qui ne soit pas d'abord punitive, mais qui suscite plutôt l'enthousiasme. Ce plan stratégique permettra également de renforcer la protection des Européens sur leur sol et de défendre mieux nos intérêts partout dans le monde. Plus de moyens pour nos armées nos gardes-frontières renforceront également la souveraineté de l'Europe et permettront à notre diplomatie d'être moins dépendante. Ce plan, enfin, permettra d'être à l'initiative d'un plan de développement économique destiné aux pays pauvres, à l'image du plan Marshall pour aider à la reconstruction de l'Europe au sortir de la guerre. Cette démarche est à entreprendre en même temps que le renforcement du contrôle des flux migratoires à nos frontières, car il est illusoire de croire que nous pouvons accueillir toute la misère du monde. Ainsi, ensemble, nous irons plus vite et plus loin. Mais ces ambitions vitales pour nos pays européens ne pourront se concrétiser que si l'Europe se dote d'un budget beaucoup plus élevé que celui de la période qui s'achève. Il devra être alimenté de plusieurs manières. Tout d'abord, par des ressources propres en lui affectant, par exemple, une part significative de la fiscalité généralisée des géants du numérique. Après la France et quelques pays européens, tous les membres de l'OCDE, États-Unis d'Amérique compris, vont enfin décider de taxer les GAFA.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la dangerosité du monde, agité par certains dirigeants aux comportements incertains et irresponsables, oblige les responsables européens à se rassembler sur l'essentiel et à ne pas être passifs et soumis au contexte international imposé par d'autres. Les bons sentiments comme une certaine naïveté n'ont que trop duré. Si nous voulons agir plus efficacement contre la pauvreté, pour un développement durable réaliste et promouvoir la démocratie partout dans le monde, l'Europe ne peut plus être celle du temps long, car les urgences nous obligent à accélérer ce temps.

doit être moins technocratique. Oui, elle doit mieux s'organiser pour concourir à armes égales dans la compétition mondiale. Oui, face à toutes les menaces, l'Europe doit continuer à renforcer la protection due à chacun de ses concitoyens. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues,

Vous m'avez aussi interrogée, tout comme le sénateur Cadic, sur l'élargissement. Je poserai quelques principes et rappellerai quelques faits. Il a toujours été admis que les Balkans occidentaux avaient une perspective européenne.

état de cause, la France parle à tout le monde. Nous recevons tous nos interlocuteurs, mais nous leur rappelons les critères à la fois internes à l'Union et externes. Vous m'avez également interrogée sur la Turquie. Dans le cadre des conclusions

Nous ne pouvons pas négocier, comme certains d'entre vous l'ont souligné, un budget de cohésion, un budget sur la PAC, c'est-à-dire des politiques qui sont extrêmement importantes pour nous, si nous ne montrons pas très activement que nous sommes ensuite capables de bien dépenser l'argent que l'Union européenne met à la disposition des acteurs au sein au sein de l'Union européenne pour soutenir des politiques publiques. Si vous voulez renforcer la position française dans ces négociations, tout ce que vous pourrez faire en tant qu'acteurs territoriaux de premier plan pour accélérer la programmation et le paiement des fonds européens dans vos territoires sera extrêmement utile. Nous pourrons ainsi montrer que, si nous négocions fortement à Bruxelles, ce n'est pas parce que nous aimons faire de grands discours, mais c'est parce que ces politiques

des discussions sur la bonne utilisation et la bonne gestion des fonds. La Cour des comptes a rendu un rapport à ce titre. Sachez que votre action dans ce domaine sera pour nous extrêmement utile.

La France souhaite poursuivre un dialogue de fermeté avec la Russie à cet égard. Les décisions de l'assemblée générale des Nations unies sur ce sujet doivent d'abord nous rappeler à la raison.

nous ne nous résoudrons pas à accepter une situation qui ne respecte pas les frontières internationalement reconnues. Les élections d'autodétermination, de souveraineté, doivent s'organiser dans un cas très précis.

Monsieur le président,madame la secrétaire d'État,mes chers collègues, permettez-moi, en conclusion de ce débat, de revenir sur l'agenda stratégique de l'Union européenne, sur lequel le Conseil européen s'est accordé pour les cinq prochaines années. Je ne rappellerai pas les quatre volets de cet agenda qui ont déjà été largement évoqués dans le débat, mais je souhaiterais souligner certaines avancées qui méritent, à mes yeux, une attention particulière. Pourquoi ? Parce que toutes témoignent d'une prise de conscience salutaire, par l'Union européenne, de la nécessité pour elle de se concevoir comme puissance, et non simplement comme espace. point, l'accent est mis par le Conseil européen sur l'importance qu'il convient d'accorder à l'euro, et plus spécifiquement au renforcement de son rôle international. La monnaie est assurément l'un des éléments fondateurs de la souveraineté. L'extraterritorialité des lois américaines, qui s'attache au dollar et contre laquelle l'agenda stratégique appelle à lutter, nous rappelle combien nous aurions à gagner à favoriser l'usage de l'euro dans les échanges internationaux. Nous pouvons aussi saluer le fait que l'agenda prévoit de finaliser l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux, sans lesquelles l'édifice de la monnaie unique reste fragile. Deuxième point : je relève une évolution sémantique sensible qui témoigne de l'éveil progressif du Conseil européen à la vision française d'une Europe-puissance. En matière de défense, l'agenda stratégique, tout en rappelant évidemment la nécessité d'une coopération étroite avec l'OTAN pour la sécurité de notre continent, invite à renforcer les moyens de la défense européenne et à viser la perspective d'une autonomie décisionnelle de l'Union européenne en ce domaine. Cet appel à l'autonomie de décision se retrouve d'ailleurs, comme en écho, dans les conclusions du sommet de la zone euro qui s'est tenu à la suite du Conseil européen. Il n'y a qu'un pas de l'autonomie à la souveraineté, qui reste néanmoins un gros mot, semble-t-il. Pourtant, le Conseil européen lui-même va jusqu'à mentionner l'impératif de souveraineté européenne dans le domaine du numérique. J'y vois la confirmation que la souveraineté numérique, à laquelle notre assemblée consacre en ce moment une commission d'enquête, est un enjeu tout à fait stratégique, qui doit se concevoir à l'échelle européenne. Troisième élément, l'agenda stratégique tel qu'il a été adopté par le Conseil européen mentionne explicitement l'impératif, pour l'Union, de se doter d'une politique industrielle. C'est un concept qui a trop longtemps été inaudible à Bruxelles, et nous pouvons nous féliciter de le voir ainsi consacré durablement. L'agenda stratégique prévoit également une mise à jour des règles européennes en matière de concurrence, que nous appelons aussi de nos voeux : il conviendra de s'assurer que cet se fasse bien au service de la stratégie industrielle que l'Union entend déployer. Enfin, quatrième motif de satisfaction : l'agenda stratégique assigne clairement à l'Union européenne la mission de développer son influence et d'être plus assertive dans la défense de ses intérêts. Il vise notamment à obtenir plus de réciprocité en matière de négociations commerciales ; c'est un objectif que nous promouvons depuis longtemps, particulièrement en ce qui concerne l'ouverture des marchés publics. Pour conclure ce débat, je veux donc saluer le nouvel agenda stratégique assigné à la Commission et au Conseil : c'est un fruit important de ce Conseil européen de 2019. Il me paraît très prometteur. Pour qu'il ne reste pas lettre morte, il doit être endossé par des personnalités qui ont à la fois l'expérience et l'ambition requises. Souhaitons donc que les prochaines nominations soient à la hauteur de cette nouvelle feuille de route de l'Union. Je formulerais un dernier souhait. L'agenda stratégique invite l'Union à consacrer plus de ressources à sa mise en oeuvre effective. Puisse en effet l'Union se doter des moyens de ses ambitions, et réveiller ainsi l'espoir d'un avenir meilleur pour l'ensemble des citoyens européens !